jours se sont écoulés depuis l'effroyable attentat terroriste qui a frappé un hussard de la République. Une fois encore, le peuple français a été touché dans sa chair. Nous ne devrons jamais oublier et nous devons réagir.

La laïcité à la française fait partie de ces valeurs républicaines qui ont forgé l'âme de notre nation et l'histoire de notre pays et que, précisément, les ennemis de la liberté veulent abattre.

Nombreux sont ceux qui souhaitent installer le doute et la division dans nos esprits. C'est ensemble que nous ferons face à la menace terroriste. Encore une fois, l'histoire exige de nous que nous soyons à la hauteur de nos responsabilités. Le chef de l'État l'a dit : « Nous ne reculerons pas.

la main de cet acte odieux : c'est l'islamisme politique, l'islamisme radical, qui n'en est pas à son premier forfait.

les ennemis de la République ont pour principal objectif de nous diviser, de faire prospérer tous les amalgames, de déchaîner la haine pour embrigader, asservir et finalement assassiner. On connaît leurs méthodes : faire le procès de la France, faire le procès de son histoire, comme si elle avait à en rougir, et de ses principes fondateurs, qui sont à l'opposé des leurs. Voilà pourquoi

On connaît aussi leurs leviers et leur mode opératoire : des lieux de culte détournés, des associations paravents et des réseaux sociaux proactifs. Comme les lâches, ils agissent dans l'ombre. l'ombre. Qu'ils sachent qu'ils trouveront toujours la République en travers de leur chemin ! Le Gouvernement, sous l'autorité du Président de la République,

la dissolution de l'une de ces associations. Très bien ! La semaine dernière, une mosquée radicale a été fermée. Qu'elle le reste ! Depuis 2018, 356 lieux de radicalisation ont également été interdits. J'ai décidé de renforcer les effectifs de renseignement, en créant cent postes dédiés à la surveillance des réseaux sociaux. Depuis le début du quinquennat, 1 250 postes supplémentaires ont été affectés à la DGSI. Vendredi dernier, je me suis rendu à Bruxelles afin de défendre auprès de la présidente de la Commission européenne et du commissaire Breton

Il n'est pas digne de renvoyer aux Français la responsabilité de cette seconde vague, car elle relève d'abord de ceux qui n'ont pas su l'analyser et agir à temps. La stratégie « tester, tracer, isoler » est un échec, et les Français n'y sont pour rien. sont pour rien. Nous attendons, ce soir, l'annonce de nouvelles mesures restrictives. Elles seront le marqueur de l'échec de notre politique de santé publique. Ayons le courage de le reconnaître

Nos champions technologiques internationaux et leurs sous-traitants ne font plus que rafistoler des poteaux tombés, en les attachant aux arbres avec de la rubalise, quand ils ne débranchent pas le voisin pour raccorder un autre. Vous allez me répondre, monsieur le secrétaire d'État, que la fibre ou toute autre possibilité de raccordement numérique sont prévues dans nos territoires d'ici à 2025, ce qui devrait tout résoudre.

voire d'un reconfinement rapide, comment nos jeunes pourront-ils continuer d'étudier et nos concitoyens avoir recours au télétravail ? Ou bien encore, comment pourrons-nous télécharger l'application

Territoires. Ma question s'adresse à M. le ministre des solidarités et de la santé. Monsieur le ministre, la crise sanitaire vous occupe, mais c'est au ministre des solidarités que je souhaite

Des milliards d'euros sont distribués aux entreprises, sans conditionnalité sociale et écologique, mais seulement quelques millions d'euros aux ménages en situation de pauvreté, alors que des mesures fiscales ont enrichi les 0,1 % des ménages les plus riches.

pour le groupe Les Indépendants -République et Territoires. Chaque année, la grippe saisonnière touche des millions de Français et entraîne des milliers d'admissions aux urgences. Le vaccin contre la grippe sauve des vies et limite les complications. Les mesures appliquées contre la covid-19 devraient ralentir la propagation de l'épidémie grippale. De façon plus certaine, il s'agit de limiter l'engorgement des hôpitaux et les erreurs de diagnostic liées à des symptômes similaires entre les deux virus. De plus, les risques de double infection semblent réels. Dans ce contexte, les Français sont très largement invités à se vacciner contre la grippe. Il en résulte une demande globale en forte augmentation. Cette année, plus de quinze millions de personnes sont destinataires de prescriptions de vaccin. Les commandes du ministère auraient été passées, en mars dernier, sur la base des chiffres de l'année précédente, augmentés de 30 %. Malgré cet effort, au-delà de la campagne de vaccination qui cible les personnes les plus vulnérables, allons-nous réellement pouvoir couvrir l'ensemble des demandes cette année ? Enfin, à la lumière de cette expérience, comment anticiperez-vous le bon approvisionnement en France des vaccins contre la covid-19 lorsqu'ils seront disponibles sur le marché mondial ?

à l'accès aux vaccins, vous pouvez compter sur le réseau des pharmaciens pour

Les Républicains. Ma question s'adresse à M. Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé. La situation épidémique de notre pays est inquiétante. L'augmentation de la circulation du virus est désormais exponentielle. Nous sommes dans la deuxième vague, et nous nous apprêtons à vivre, malheureusement, le de la précédente. La première vague a été celle de l'improvisation : ni masque, ni gel hydroalcoolique, ni blouses

Aux discours contradictoires de l'exécutif, se sont malheureusement ajoutés ceux, tout aussi contradictoires, des scientifiques, éblouis pour certains par les feux de la rampe. La seconde vague est celle de l'impréparation.

missionné par le Premier ministre en avril dernier, a proposé vingt et une solutions pour mieux gérer la crise sanitaire. Le minimum aurait été d'en informer le Parlement ou, au moins, la commission d'enquête, ce qui n'a pas été le cas. Le répit laissé par le virus, cet été, aurait dû être mis à profit pour mieux nous préparer. Il n'en a rien été. On a laissé les Français se faire tester en masse, pour faire du chiffre, sans stratégie, ce qui a embolisé le système avec des résultats qui mettaient parfois plus d'une semaine à arriver. Si l'on a beaucoup parlé des brigades sanitaires, peu les ont vues. Pourquoi ne pas avoir mis à profit ce mois d'été pour préparer l'ouverture de lits de réanimation supplémentaires ? Vous en avez annoncé 12 000 le 27 août dernier ; il n'y en a que 5 700, dont 5 000 sont opérationnels. Veuillez poser votre question ! ... des étudiants, des aides-soignants, des infirmiers, des internes pour venir en renfort dans les services de réanimation en tant que de besoin ? Ma question, monsieur le ministre, est simple : espérez-vous sortir un jour la France de cette crise ?

cet été, plusieurs milliers de soignants ont été formés, non pas par le Gouvernement ni par vous, d'ailleurs, mais par les hôpitaux, les facultés, les régions, dont l'action a été déterminante, augmentant les capacités de formation exprès de plusieurs milliers de soignants pour qu'ils puissent participer aux soins dans les services de réanimation. 15 % de lits de réanimation supplémentaires ont été ouverts de façon pérenne dans notre pays. Vous pouvez considérer que c'est peu, mais, pour les hôpitaux qui ont fait cet effort en trois mois, je peux vous garantir que c'est beaucoup ! Monsieur le sénateur Milon, vos chiffres datent

la réouverture des discothèques à Marseille, des restaurants à Lyon ou encore des bars à Saint-Étienne, à telle enseigne qu'une seconde délibération a été demandée dans l'urgence par les sénateurs, voyant l'erreur qui avait été commise. C'est faux ! Menteur ! La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour le groupe Union Centriste.

Mais, depuis quelques jours, des attaques d'une violence inacceptable contre le Président de la République et contre la France se propagent des médias des pays arabes et des médias turcs, qui sont autant de vecteurs de haine, pouvant inciter à la violence physique. Tour Eiffel ensanglantée, discours haineux ou gravement antisémites, appels à la violence ... La chaîne qatarienne Al-Jazeera en arabe multiplie les attaques, comme la chaîne turque TRT. On sait que le Qatar et la Turquie soutiennent la mouvance des Frères musulmans, dont j'ai demandé à de multiples reprises l'interdiction en France. Leur leader Youssef Al-Qaradawi, interdit de séjour dans de nombreux pays européens, multiplie les appels à la haine. L'un des derniers en date était un hommage appuyé au travail d'Hitler, dans lequel il précisait que, même en chaise roulante, il irait

particulièrement vigilant pour réprimer l'incitation à la haine, à la violence ou d'autres manquements. Il y a dix ans, le CSA avait interdit la chaîne du Hamas, Al-Aqsa, et même la chaîne Al-Manar. Or la situation, en 2010, était bien moins grave que celle que nous connaissons aujourd'hui. Dès lors, ma question est simple, monsieur le ministre : allez-vous engager des procédures pour interdire la chaîne Al-Jazeera et la chaîne TRT des réseaux français ? La

République a déclaré vouloir couper les influences étrangères des affaires intérieures françaises était juste : en France, nous considérons que les Français de confession musulmane ne relèvent d'aucune puissance étrangère.

Celles-ci vous ont adressé une demande claire, unanime : le retrait définitif de votre réforme de l'assurance chômage. Cette réforme n'a qu'un but économiser sur l'indemnisation du chômage. C'était déjà terriblement injuste, mais, devant le drame économique qui se joue, c'est indigne, c'est inhumain et c'est contraire à l'avenir des forces du travail, qu'il faut préserver. C'est tellement vrai que vous n'osez pas appliquer cette réforme. Vous l'avez reportée de trois mois une première fois, puis maintenant une seconde fois. Mais vous persistez à vouloir l'appliquer plus tard. Pourquoi cet entêtement ? Des centaines de milliers d'emplois vont être détruits, menacés, fragilisés par la crise. On annonce près de 1,2 million de chômeurs supplémentaires l'année prochaine. Appliquer cette réforme aujourd'hui serait un scandale, parce que c'est l'inverse de ce qu'il faut plus de protection sociale, et non pas moins ! Le plan de relance donne beaucoup d'argent aux entreprises, mais le Medef continue de demander des économies sur le chômage. C'est inacceptable. Ma question est simple, madame la ministre : pourquoi refusez-vous d'entendre l'évidence ? Qu'attendez-vous pour abandonner cette réforme ?

la conférence du dialogue social organisée par le Premier ministre avec les partenaires sociaux. Compte tenu de la situation sanitaire, il existe aujourd'hui un consensus pour reporter l'application de cette réforme. Le Gouvernement fait pleinement confiance au dialogue social et aux partenaires sociaux pour trouver de nouveaux équilibres. Il est prêt à adapter des paramètres à la nouvelle situation de l'emploi. Pour autant, permettez-moi de vous le

que nous agissons depuis le début de la crise pour protéger tous les salariés et toutes les compétences. Nous avons mis en place en avril dernier un dispositif d'activité partielle d'une ampleur inédite, lequel a permis de préserver l'emploi de près de 9 millions de Françaises et de Français. Vous y croyez ? Monsieur le sénateur,

Elle permettrait d'économiser 1,5 milliard d'euros en 2021 et 2,6 milliards d'euros en 2022. On donne 100 milliards d'euros au plan de relance et on n'a qu'une obsession : économiser 2,5 milliards en 2022 sur le dos des chômeurs

Républicains. Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Depuis des mois, la Turquie de M. Erdogan multiplie les provocations à l'égard de ses alliés occidentaux chantage aux flux migratoires, achat d'armes russes pour fragiliser l'OTAN, forages gaziers illégaux dans les eaux grecques et chypriotes, offensives contre nos alliés kurdes en Syrie, ingérence en Libye. Pis encore, de manière irresponsable, au lieu d'agir en faveur de la paix, la Turquie attise le terrible conflit du Haut-Karabakh en envoyant des avions, des drones suicides et des mercenaires pour soutenir l'offensive de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Cela n'est pas encore suffisant. Alors que la France vient de traverser un drame épouvantable, le président turc offense, par ses propos, le Président de la République, insultant par là même notre pays, tout entier. comble de l'inacceptable est cet amalgame inadmissible avec la situation des juifs dans les années trente, qui donne la nausée. Monsieur le ministre, va-t-on une fois de plus et sans réagir supporter longtemps d'être le bouc émissaire de la crise économique et politique qui secoue la Turquie ?

Connaissez-vous, monsieur le ministre, un banquier qui prête de l'argent pour se faire copieusement insulter ? La France, nous dit-on, a, comme ses voisins, des intérêts économiques en Turquie. Je ne les méconnais pas, mais l'appel au boycott des produits français est déjà une réponse qui devrait nous inciter à beaucoup plus de lucidité sur l'avenir de nos entreprises dans ce pays. Ma question est bien simple : quelles mesures allez-vous prendre, au niveau national comme au Conseil européen de décembre prochain, où le soutien mou, ... Il faut conclure. ... pour sanctionner ce dirigeant nationaliste qui veut jouer à l'empereur ottoman, alors qu'il fait offense à son peuple et à l'histoire même de la Turquie

Je crois que nous avons été le fer de lance de cette prise de conscience européenne, qui, vous avez raison, n'est pas encore suffisante. Cependant, les mots de solidarité qui ont été exprimés sans ambiguïté ces derniers jours par l'ensemble des dirigeants européens sont aussi un fait nouveau, qui marque l'évolution du consensus vers la position de fermeté qu'a défendue la France. Nous irons plus loin. Nous continuerons cette stratégie de réactions françaises et européennes. Cela peut passer par de nouvelles sanctions. Je rappelle que la France en avait déjà pris l'initiative l'an dernier, après les forages dans les eaux chypriotes. Nous avons un rendez-vous au Conseil européen de décembre : nous pousserons évidemment en faveur de mesures européennes fortes, dont la possibilité de sanctions. Il faut être précis : cela ne doit pas être le résumé de notre politique étrangère, y compris à l'égard de la Turquie.

La deuxième vague et les mesures qui vont être prises dans les prochaines heures vont encore prolonger les terribles effets de ces restrictions pour beaucoup de Français. Ainsi, 1 million de Français sous le seuil de pauvreté ont rejoint les plus de 9 millions qui y étaient déjà, chiffre en augmentation depuis 2018. cette situation dramatique, il aurait fallu réagir plus en amont, plus rapidement et plus efficacement. Vos annonces de samedi dernier ne répondent pas à ces trois impératifs. Vous pratiquez un saupoudrage qui ne prend pas en compte l'ampleur de ce qui est déjà là et encore moins de ce qui attend notre pays. Votre plan est centré sur l'insertion par l'activité : cela est certes nécessaire, mais insuffisant, en particulier compte tenu des perspectives de créations d'emplois qui sont celles d'aujourd'hui. Les jeunes les plus précaires, les nouveaux précaires sont sortis de vos radars. À ceux-là, vous proposez des aides exceptionnelles et ponctuelles, quand la deuxième vague nous confirme qu'un grand nombre de Français risquent de s'installer dans une précarité sur un temps long. Il faut donc ouvrir le revenu minimum aux jeunes pour les empêcher de sombrer, revenir sur votre réforme des aides personnalisées au logement, revaloriser les minima sociaux, augmenter la part du plan de relance pour soutenir les plus précaires, notamment en ce qui concerne l'aide alimentaire. Les associations caritatives nous ont dit que cette demande explosait depuis six mois. Elle a parfois été multipliée par deux, voire par trois. Ne nous répondez pas qu'il ne faut pas laisser les populations stagner dans les minima sociaux : la question n'est plus là. La seule qui doit se poser est la suivante allez-vous enfin adapter votre politique de lutte contre la pauvreté à la situation actuelle ?

pour ne laisser personne sur le bord de la route. C'est pourquoi nous augmentons de nouveau le nombre de places en insertion par l'activité économique (IAE) : aux 100 000 places prévues s'ajouteront 30 000 places supplémentaires, comme l'a annoncé le Premier ministre. Le budget pour 2021 prévoyait déjà 1,2 milliard d'euros pour l'IAE, soit 204 millions de plus qu'en 2020. Samedi, le Premier ministre a annoncé 150 millions d'euros supplémentaires pour l'IAE. C'est inédit et essentiel. L'insertion par l'activité économique sera l'une des clés pour lutter contre le chômage, donc pour lutter contre la précarité. Madame la sénatrice, nous entendons l'urgence sociale et économique. C'est pourquoi nous avons reporté la réforme de l'assurance chômage de trois mois. Je répète que cette réforme réforme est une bonne réforme, mais elle doit être adaptée à la situation. Le Gouvernement s'est donc donné trois mois supplémentaires pour dialoguer avec les partenaires sociaux. Certains paramètres Certains paramètres vont être adaptés. Plus précisément, le contexte sanitaire et économique a mis en lumière les difficultés pour les personnes en contrat court. en contrat court. Un nombre important de salariés précaires qui parvenaient, avant la crise, à enchaîner suffisamment de contrats courts pour maintenir un certain niveau de revenus ne le peuvent plus. Il s'agit des saisonniers, des extras de l'hôtellerie et de la restauration ou de l'événementiel, mais pas seulement. Nous sommes très attentifs à leur situation et cherchons actuellement des solutions. Madame la sénatrice, vous le comprenez, nous ne laisserons personne sur le bord du chemin. Madame la ministre, votre réponse est pour le moins très évasive

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur. Le 18 octobre dernier, le conseil de défense a annoncé que 231 personnes étrangères en situation irrégulière et soupçonnées de radicalisation seraient reconduites dans leur pays d'origine. Au-delà de leur cas particulier se pose la question de l'efficacité de notre système en matière de retour dans les pays d'origine des personnes étrangères en situation irrégulière sur notre territoire.

que l'on puisse travailler sur ce sujet, car, si nous n'obtenons pas de laissez-passer consulaires dans de bonnes conditions de la part des pays sources, nous n'y arriverons

La parole est à M. Philippe Folliot, pour le groupe Union Centriste. Madame la ministre de la défense, depuis quelques mois, la multiplication de comportements inamicaux, voire agressifs de la Turquie envers ses alliés de l'OTAN en général et de la France en particulier pose un grave problème. L'incident avec la frégate, au mépris des règles de l'Alliance, les explorations sauvages en Méditerranée orientale, au mépris du droit de la mer, la livraison d'armes à la Libye, au mépris de l'embargo décidé par l'ONU, l'intervention au Haut-Karabakh, au mépris des équilibres régionaux, et, pour finir, les insultes contre le président Macron, au mépris des usages diplomatiques les plus élémentaires : tout cela fait beaucoup, tout cela est trop Le peuple turc ne saurait être assimilé aux outrances d'un président confronté à une contestation populaire majeure, les lourdes défaites électorales récentes agitant, avec l'énergie du désespoir, un islamisme conservateur et agressif. Un des symboles en est le sabordage de l'héritage du moderniste et visionnaire Mustafa Kemal, dit « Atatürk », notamment au travers de la transformation de Sainte-Sophie de musée en mosquée. Nous avons régulièrement abordé ces questions et ces différends au sein de l'assemblée parlementaire de l'OTAN, en relevant notamment que le président turc ne se comportait pas comme un allié respectueux de nombre de principes démocratiques et ignorait les articles fondateurs 4 et 5 du traité de l'Alliance. Quelle réponse apportez-vous au décalage entre les actes du président populiste Erdogan et les obligations qui lui incombent en tant qu'allié de la France au sein de l'OTAN ? Madame la ministre, selon vous, la Turquie peut-elle et doit-elle rester dans l'OTAN ?

la Turquie a adhéré à l'OTAN en 1952 et a apporté, pendant de nombreuses années, sa contribution à la sécurité euro-atlantique.

le fait même que la Grèce et la Turquie appartiennent à la même alliance a pu contribuer à apaiser certaines tensions entre ces deux pays. Mais, depuis quelques mois, nous assistons à une situation tout à fait inédite où la Turquie pratique la politique du fait accompli

Le constat que je dresse est celui d'un allié qui ne se comporte pas en allié. Face à cette situation, il n'est qu'une seule attitude possible : rappeler à la Turquie les obligations qui s'imposent à elle en tant qu'alliée.

La fermeture partielle ou totale des cafés, des débits de boissons, des restaurants ou encore des hôtels, en raison du manque de clients, est une mesure qui concerne de plus en plus de territoires. L'explosion du nombre de contaminations de ces derniers jours nous permet de douter de l'efficacité de ces mesures. En dépit des protocoles sanitaires, la question du reconfinement refait surface. Lors de la première vague, le Gouvernement s'est montré assez réactif sur la prise de mesures compensatoires à l'arrêt d'activité des établissements recevant du public, tels les hôtels ou encore les bars et restaurants. Toutefois, le défi est aujourd'hui tout autre : alors que nous entrons dans une seconde vague, sans doute plus violente et plus longue, les professionnels du tourisme ne peuvent se satisfaire de mesures compensatoires et doivent se voir proposer un véritable horizon. Le Gouvernement a présenté un plan France Relance qui prétend « faire la France de demain ». Or, faire la France de demain, c'est s'appuyer sur ses forces, et notamment sur ses territoires. Le tourisme est une de ces forces : les professionnels de ce secteur offrent des emplois durables, non délocalisables. Ce sont également des savoir-faire que le monde entier nous envie. Il faut penser à demain. Un jour nous vaincrons ce virus ; en attendant, nous devons préserver la filière du tourisme et de l'hôtellerie-restauration. Aussi, et avant les nouvelles annonces de ce soir, pourriez-vous nous préciser ce que le Gouvernement prévoit pour permettre à ces métiers, qui mettent en valeur nos territoires, de s'adapter concrètement aux mesures imposées par la situation sanitaire ? ? Comme vous le savez, dès avant la crise sanitaire, la filière hôtellerie-restauration peinait à recruter. Pourquoi ne pas faire de cette période troublée une opportunité pour favoriser la formation de nos jeunes à ces nombreux métiers, par des dispositifs innovants de formation à distance ou en présentiel, dans les établissements hôteliers et de restauration désormais fermés au public ? Monsieur le ministre, nous nous devons d'anticiper l'avenir pour préserver cette filière particulièrement touchée par la crise sanitaire.

raison pour laquelle l'ensemble du ministère de l'économie, des finances et de la relance est mobilisé pour soutenir les secteurs les plus fragilisés, notamment celui des cafés, hôtels et restaurants (CHR) et ceux qui en dépendent.

Le 14 juillet, le Président de la République disait : « Nous serons prêts pour une deuxième vague ». Vous nous permettrez aujourd'hui, en attendant les annonces de ce soir et en soulignant la précipitation, la mise en scène et la dramaturgie qui les entourent dans la presse, de douter de cette affirmation du 14 juillet.

vous maîtrisez le verbe, vous nous parlez avec énergie ... On a même souvent un peu d'empathie pour vous, car vous faites un job qui n'est pas facile. Mais cette habileté est aussi faite de beaucoup de semi-vérités : semi-vérité sur les tests, semi-vérité sur la stratégie d'isolement, semi-vérité sur les lits de réanimation- vous en annonciez 14 000, je pense que nous serons plus

responsable et mature. Quand allez-vous sortir de la posture politique, voire politicienne, pour leur parler à la hauteur de ce qu'ils sont ?

Madame la sénatrice, comme j'aurais aimé que surgissent de votre question une idée, une proposition ou même une orientation générale à laquelle ni la France, ni l'Europe, ni les États-Unis n'auraient songé pour lutter contre la pandémie la plus meurtrière de notre histoire contemporaine !

vous vous livrez à une nouvelle attaque en piqué. En fait, vous n'avez rien à dire ! Madame la sénatrice, on ne sauve pas des vies avec des attaques politiques ; on ne soutient pas les soignants avec des attaques politiques ; on n'encourage pas les Français à tenir bon dans cette période difficile avec des attaques politiques.

l'épidémie de la covid-19 est incontrôlée et la situation dans nos hôpitaux devient très périlleuse. Certains services de réanimation sont d'ores et déjà saturés. L'épidémie flambe et des Français meurent. Votre devoir, monsieur le ministre, est non seulement de protéger à tout prix les Français, mais aussi et avant tout d'anticiper. Le Conseil scientifique avait prévu dès juillet dernier une deuxième vague. Aujourd'hui, cette vague déferle, incontrôlée, et les Français ont le sentiment que rien n'a été anticipé depuis la fin du confinement, que rien n'a changé à l'hôpital par rapport au printemps Il est vrai que l'organisation hospitalière aurait mérité qu'un plan d'anticipation soit élaboré pendant l'été afin de pouvoir augmenter rapidement le nombre de soignants et permettre l'ouverture d'un plus grand nombre de lits de réanimation. Monsieur le ministre, plutôt que de dévaloriser certaines professions paramédicales en accordant des autorisations temporaires d'exercice à des personnes qui n'ont pas d'expérience, pourquoi ne pas s'autoriser à surclasser, un temps de formation, et pour quelques tâches limitées, les aides-soignants et les infirmiers, comme l'a suggéré le professeur Philippe Juvin, chef du service des urgences de l'hôpital européen Georges-Pompidou à Paris ? Paris ? La parole est à M. le ministre des solidarités et de la santé. Pour le coup, madame la sénatrice Drexler, vous avez parfaitement raison : il faut anticiper et être capable de former davantage de personnels soignants.

Quels en sont les enjeux ? Il s'agit d'abord du maintien, voire du renforcement, d'un tissu d'agriculteurs maillant notre pays, vivant de leur production, assurant le socle de notre ruralité et donc de notre pays. ensuite d'assurer la souveraineté alimentaire de la France et une alimentation saine. Il s'agit enfin de répondre aux évolutions climatiques et environnementales, à la préservation du vivant. L'accompagnement des mutations à opérer pour s'engager dans une agriculture plus durable, plus raisonnée, est essentiel. Il ne doit pénaliser ni ceux qui sont déjà engagés sur ce chemin, bien contraire, ni ceux qui amorcent cette transformation qu'il faut encourager et protéger, sans jamais oublier l'objectif premier d'indépendance alimentaire. Je pense en particulier aux zones de montagne, où les efforts déjà accomplis seront, je l'espère, reconnus. Avec cette nouvelle PAC et les 62 milliards d'euros que la France touchera, nous nous engagerons dans un véritable changement de paradigme avec l'obligation de pratiques agronomiques exigeantes comme socle du futur régime d'aides et l'ajout d'écorégimes nationaux pour ceux qui iront au-delà des minima légaux exigibles. Il apparaît donc essentiel de poursuivre la recherche d'un double équilibre : celui de la cohérence européenne et celui de la reconnaissance de la diversité et de la richesse agricole de la France au titre du plan stratégique quelle garantie avons-nous de ne pas aboutir à vingt-sept politiques agricoles nationales divergentes, mais au contraire d'aller vers une convergence des normes ? Quelle différenciation territoriale intégrera le futur plan stratégique national ?

tous les États membres. Nous avons obtenu là une très grande avancée pour nos agriculteurs. Enfin, je terminerai en posant une simple question : quel secteur d'activité

La séance est reprise. Mes chers collègues, pour le respect des règles sanitaires, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dans l'hémicycle, y compris pour les orateurs. Il vous est demandé de laisser un siège vide entre deux sièges occupés. J'invite chacune et chacun à veiller au respect des distances de sécurité. Je rappelle également que les sorties de la salle des séances devront exclusivement s'effectuer par les portes situées au pourtour de l'hémicycle. Mes chers collègues, les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie ce jour sont consultables sur le site du Sénat. En l'absence d'observations, je les considère comme adoptées.- Questions J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » est parvenue à l'adoption d'un texte commun. J'informe le Sénat que les candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire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

1 du projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières. Tous ceux qui ont voté pour, à l'exception de MM. Philippe Bonnecarrère et Bernard Delcros, de Mme Annick Jacquemet, et de M. Jean-François Longeot, voulaient en réalité voter contre. Tous ceux qui ont voté contre souhaitaient voter pour

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement

Monsieur le président, monsieur le président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, madame la rapporteure, messieurs les rapporteurs pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, la France est une grande nation scientifique, nous ne le répéterons jamais assez. Au-delà des formules convenues, nous parlons d'un patrimoine qui nous a été transmis et qui nous permet de nous projeter vers notre avenir commun. La République a noué un pacte avec ses scientifiques, ses chercheurs, ses enseignants-chercheurs, ainsi qu'avec les institutions qui travaillent chaque jour à repousser les frontières de notre ignorance. Je songe évidemment à nos universités, nos écoles et nos organismes de recherche. La III République a été la première à reconnaître la liberté académique dans les universités et à donner toute leur place aux professeurs. Elle a jeté les fondements, avec le CNRS, de la création de nos grands organismes de recherche nationaux, qui se sont ensuite développés tout au long des dernières décennies. C'est toujours dans les moments de grands défis nationaux de reconstruction et face à l'adversité la plus immédiate que se manifeste la relation particulière qui s'est nouée depuis près de deux siècles entre la science et les institutions républicaines. Il n'est pas nécessaire de rappeler la contribution immense de nos scientifiques à la reconstruction de notre pays après la guerre. L'actualité suffit à le démontrer : nos chercheurs et nos enseignants-chercheurs sont montés en première ligne face à la covid-19. Le rapport du groupe de travail de votre commission de la culture l'a très justement établi.

se sont mobilisés pour contenir l'épidémie, trouver des traitements, tester des vaccins, évaluer l'impact social de la crise. Plus récemment encore, l'ensemble du monde scientifique s'est joint, dans le sillage du Président de la République, à l'hommage rendu la semaine dernière à Samuel Paty, à la suite de l'attentat abject de Conflans-Sainte-Honorine. Au-delà des hommages, chacun dans cet hémicycle mesure à quel point nous aurons besoin de nos universitaires et de nos chercheurs pour mieux comprendre les ressorts et les causes des radicalités, notamment islamistes, qui ont trop souvent frappé notre pays depuis déjà de trop nombreuses années. Chacun le comprend, nous devrons mobiliser, plus que jamais, toutes nos forces de recherche, particulièrement dans le domaine des sciences humaines et sociales, pour nous donner les leviers de compréhension et d'action face à la menace terroriste. Notre République s'est nourrie des travaux de ses sociologues, de ses historiens, de ses juristes, bref de tous ceux qui nous permettent de comprendre notre monde, et elle s'en nourrira encore. Le projet de loi que j'ai l'honneur de défendre devant la Haute Assemblée a été annoncé voilà un peu plus de dix-huit mois, le 1 février 2019, dans le cadre de la célébration des 80 ans du CNRS. Le travail de préparation de ce texte a été long. Il a été nourri d'une large consultation et de près d'un millier de contributions. Il a été scandé par les travaux de plusieurs groupes de travail. Il a surtout été inspiré par des centaines de déplacements et de rencontres que j'ai pu faire, au plus près du terrain, au plus près de nos chercheurs, dans les laboratoires, au coeur des universités et des organismes, et ce partout en France. Au-delà des postures politiques, ce qui s'est exprimé chaque fois, c'est un besoin manifeste : nos scientifiques nous demandent plus de temps, plus de moyens et plus de visibilité dans leur travail. Ils nous demandent plus de considération et peut-être une meilleure écoute, particulièrement en temps de crise. Le projet de loi que je vous soumets aujourd'hui vient renouveler et ancrer dans la durée ce pacte entre la Nation et la connaissance, entre la Nation et sa recherche, entre la Nation et ses chercheurs. Car c'est à eux que cette programmation s'adresse d'abord, et les centaines de visites que j'ai effectuées depuis trois ans pour aller à leur rencontre dans les laboratoires m'ont convaincue que nous avons à leur égard un devoir de vérité. Il est grand temps de dire certaines réalités sans langue de bois. Oui, la recherche française décroche progressivement du top 10 mondial, comme en témoigne sa rétrogradation du cinquième au huitième rang en matière de publications scientifiques. Non, il n'est pas décent qu'à bac+8, après plusieurs années de postdoctorat, un jeune chercheur soit recruté à 34 ans pour un salaire équivalent à 1,4 SMIC. Non, une grande agence nationale de financements ne peut pas écarter plus de 80 % des projets qui lui sont soumis. Oui, l'attractivité de la recherche française est en péril, et le parcours de notre dernier prix Nobel de chimie, Emmanuelle Charpentier, qui, après avoir obtenu son doctorat en France, a effectué tout le reste de sa carrière à l'étranger, est emblématique d'une fuite des cerveaux qu'il nous faut impérativement juguler. Cette page de notre histoire scientifique ne fait ni justice à notre recherche ni honneur à notre pays, et nous devons la tourner pour de bon. Pour autant, la suivante ne sera pas vierge. Dire la vérité, ce n'est pas seulement regarder le verre à moitié vide, c'est aussi mesurer nos forces. Le prix Nobel d'Emmanuelle Charpentier n'évoque pas seulement notre difficulté à retenir nos talents, il nous parle aussi de l'excellence de notre enseignement supérieur et de nos formations. Et ce n'est pas là notre seul atout Je pense à nos UMR, les unités mixtes de recherche, à nos instruments et à nos infrastructures de recherche, et, bien sûr et avant tout, à nos chercheurs, nos enseignants-chercheurs, nos ingénieurs, nos techniciens, nos personnels de soutien, qui sont notre plus grande richesse, parce qu'ils ont des idées plein la tête, parce qu'ils ont de l'or dans les mains, parce qu'ils ont en eux le feu sacré du pionnier, de l'« arpenteur de l'infini », pour reprendre une image chère au mathématicien Alexandre Grothendieck. L'extraordinaire engagement dont ils font preuve depuis le mois de mars l'illustre magnifiquement. Grâce à ce terreau d'exception, notre pays est encore capable d'attirer des scientifiques de renommée internationale. L'an dernier, l'Université de Strasbourg a fait venir à l'Institut de sciences et d'ingénierie supramoléculaires le chercheur américain Richard Schrock, prix Nobel de chimie en 2005. Cette année, ce sont Esther Duflo et Abhijit Banerjee, tous deux prix Nobel d'économie, qui reviennent enseigner en France, à l'École d'économie de Paris et à l'Université Paris Sciences & Lettres. C'est bien la preuve que, lorsque nous nous en donnons les moyens, nous pouvons convaincre les meilleurs de rejoindre nos établissements. Par conséquent, il est grand temps de capitaliser sur nos forces scientifiques, en nous attaquant à la racine du mal plutôt qu'à l'efflorescence de ses symptômes. Le sous-investissement chronique dans notre recherche est tel que l'on peut parler d'une décennie perdue. L'objectif de consacrer 3 % de notre PIB à la recherche, affiché voilà vingt ans dans le cadre du traité de Lisbonne, n'a jamais été atteint. Il est devenu le symbole de notre incapacité collective à tenir nos engagements envers la communauté scientifique. C'est là la source du sentiment de malaise, de défiance et parfois de colère qui couve dans nos laboratoires. Ces années de promesses non tenues, de livres blancs sans lendemain et de réformes de structure sans effet sur un quotidien qui n'a cessé de se dégrader nous obligent à l'égard de la communauté scientifique. Nous leur devons un horizon, une ambition forte et le chemin pour l'atteindre. La programmation que je vous soumets aujourd'hui est celle qui, pour la première fois depuis des décennies, changera la donne pour nos chercheurs, parce que c'est une programmation du réel, une programmation soutenable, atteignable, ancrée dans notre réalité budgétaire, nationale et européenne. C'est cette vérité-là, cette sincérité-là, que nous leur devons par-dessus tout. Cette programmation construit, marche après marche, le socle de notre politique de recherche. L'investissement de 25 milliards d'euros qu'elle porte conduira à augmenter de 20 % les moyens de la recherche et sanctuarisera son budget à hauteur de 20 milliards d'euros en 2030.

timide. C'est la durée nécessaire à la mise en place progressive des moyens et des outils qui les accompagnent, c'est l'horizon 2030 fixé par les Nations unies en faveur du développement durable. C'est enfin une durée sécurisée par une clause de revoyure, dont la première marche est consacrée par le projet de loi de finances pour 2021, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale ce lundi à une large majorité. Cette première marche, consacrée par le projet de loi de finances, est raffermie grâce aux financements du plan de relance, qui créent le choc budgétaire de début de période que nombre d'entre vous appellent de leurs voeux. Mais ce budget cible est un budget plancher : il ne résume pas à lui seul tous les moyens dont bénéficiera la recherche durant les prochaines années. La programmation est en effet le vaisseau amiral d'une entreprise globale de soutien à la recherche française, qui s'alimentera à d'autres sources le quatrième plan d'investissements d'avenir, la nouvelle génération de contrats de plan État-région (CPER) et le neuvième programme-cadre de recherche et d'innovation européen se présentent dans le même calendrier que ce projet de loi. Cette synchronisation des horloges n'a rien de fortuit et donne tout son sens à la durée de cette programmation : dix ans, ce n'est pas seulement la temporalité d'un projet de recherche, c'est l'amplitude du programme Horizon Europe, la préparation et le début, toujours important, du programme qui le suivra, c'est la succession de deux vagues de CPER, c'est le temps de la respiration de la recherche elle-même, qui est différent du temps institutionnel et que nous devons prendre en compte en tant que tel. Grâce à cette synergie de moyens, la prochaine décennie sera celle du renouveau de notre recherche. Dans les deux prochaines années, plus de 6,5 milliards d'euros seront consacrés, dans le plan de relance, à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. La place faite à la science dans notre réponse à la crise, c'est la promesse d'une relance durable et ambitieuse, qui ne se contentera pas de reprendre notre économie là où on l'avait laissée ou de reconduire à l'identique l'existant. Elle transformera cette crise, qui deviendra une opportunité de bâtir une société écologique, solidaire et souveraine, grâce à l'intelligence, à l'inspiration, à l'innovation en germe dans nos laboratoires et nos amphithéâtres. La programmation de la recherche dans le cadre de ce projet de loi permettra ainsi de nous doter, sur le modèle des lois de programmation militaire et de leur réexamen périodique, d'un cadre d'actualisation régulier, qui permettra au Parlement de se prononcer, au moins tous les trois ans, sur les leviers mis à la disposition de notre recherche publique comme privée. Ce que propose Ce que propose ce projet de loi, c'est non pas un panel de réponses définitives pour les dix prochaines années, mais un chemin qui permettra aux gouvernements et aux majorités parlementaires à venir de se prononcer sur leurs ambitions pour notre communauté scientifique. C'est bien l'ambition de construire une programmation sur le temps long. Cette ambition repose sur quatre convictions, qui forment les quatre axes de la programmation que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. La première de ces convictions, c'est que la recherche forme un seul et même continent, dont tous les territoires doivent être correctement irrigués si nous voulons résoudre les énigmes de notre temps. C'est pourquoi ce projet de loi programme un réinvestissement inédit et massif dans tous les domaines de la connaissance. La physique de l'atmosphère ne relèvera pas seule le défi du réchauffement climatique ; l'histoire de l'art ne pansera pas seule les blessures de la cathédrale Notre-Dame la biologie seule ne suffira pas à enrayer la crise sanitaire. L'une aura besoin de la glaciologie, de la chimie, de la sociologie, de l'économie, l'autre de la physique des matériaux, de l'archéologie et de la musicologie, et, la dernière, de la zoologie, de la psychologie et des sciences informatiques. Face à l'inconnu, non seulement nous avons besoin de science, mais nous avons besoin de toute la science, qu'elle soit exacte, humaine ou sociale. Car les défis contemporains surgissent précisément au carrefour des disciplines et exigent d'être approchés globalement. C'est pour prendre acte de cette complexité que nous avons fait le choix d'une programmation transversale, non fléchée, dénuée d'sectoriel, mais néanmoins attentive à couvrir les besoins de toutes les disciplines. Notre agence nationale de recherche est le pivot de cette stratégie. L'augmentation de son budget à hauteur de 1 milliard d'euros répond à une ambition majeure : l'ouverture. Nous devons ouvrir ses financements à toutes les disciplines, à toutes les démarches, qu'elles soient purement exploratoires ou en prise directe avec les priorités du pays, à tous les laboratoires, ceux des organismes et des grandes universités pluridisciplinaires comme ceux des universités à la signature territoriale affirmée, grâce à un taux de succès de 30 %, contre 16 % aujourd'hui, conforme aux standards internationaux. Nous devons ouvrir ces financements au-delà même des équipes lauréates, grâce à un préciput à hauteur de 40 %, qui permettra d'alimenter les projets des autres équipes, de leurs laboratoires et de leurs établissements de tutelle, tous partenaires de leur réussite. de la recherche (ANR) de renouer avec sa vocation universelle, en faisant voler en éclat les vieux clivages entre les sciences exactes et les sciences humaines et sociales, entre la recherche appliquée et la recherche fondamentale, entre le financement sur projet et le financement récurrent. par le biais du préciput, ce ne sont pas moins de 450 millions de crédits de base qui viendront irriguer tous les territoires, scientifiques et géographiques. À ces moyens inédits s'ajoutera, dès 2021, une hausse de 10 % des moyens des laboratoires dès 2021 et, à l'horizon 2023, %. J'aurai l'occasion de vous présenter des amendements non seulement pour apporter des clarifications sur la question du préciput, mais également pour prendre acte, dans la loi, de mon souhait de renforcer les moyens de base des laboratoires. de base des laboratoires. Notre recherche ne souffre pas d'un excès de financement par appel à projets : notre recherche souffre d'un défaut de financement global, de base et par appel à projets. L'ambition de ce projet de loi, c'est non pas de favoriser l'un par rapport à l'autre, mais bien de travailler à renforcer l'ensemble des canaux de financement de la recherche. la montée en puissance de l'ANR prend acte de la dimension foncièrement collective de l'entreprise scientifique. Cette préoccupation est en réalité le fil rouge de l'ensemble du texte. Il affleure tout particulièrement dans le deuxième axe de la programmation : il s'agit de faire émerger une nouvelle génération de scientifiques, en redonnant aux carrières la reconnaissance et l'attractivité qu'elles méritent.

la rémunération, les moyens et les opportunités qui leur sont donnés ne sont pas à la hauteur de leur travail, et bien loin d'attirer les jeunes qui pourraient leur succéder. La compétition pour les talents est devenue internationale et on ne peut prétendre rivaliser avec des salaires dérisoires et des débuts de carrière laborieux. Afin de combler ce fossé, la programmation engage un véritable choc d'attractivité des carrières scientifiques, et ce dès le doctorat, car il est grand temps de redonner toutes ses lettres de noblesse à notre troisième cycle. Ainsi, le nombre de contrats doctoraux financés par le ministère sera augmenté de 20 %, avec l'objectif de ne laisser aucun doctorant sans salaire, et en portant une attention particulière aux thèses en sciences humaines et sociales, dont moins de 40 % font actuellement l'objet d'un contrat. Leur financement sera par ailleurs rehaussé de 30 % d'ici à 2023. Pour sécuriser la transition vers un poste pérenne, la programmation prévoit également de créer un contrat postdoctoral public ou privé. Au-delà des premiers pas dans la recherche, ce sont les prémices de la carrière scientifique qui doivent être soutenues. Le salaire d'entrée des jeunes chercheurs est devenu le symbole de la dévalorisation de notre recherche et c'est la raison pour laquelle je me suis engagée très tôt à ce qu'aucun maître de conférences ou chargé de recherche ne soit plus recruté au-dessous d'un salaire équivalent à deux SMIC. Cette promesse sera tenue dès 2021. Bien entendu, afin de ne pas créer d'inversion de carrière, les maîtres de conférences et les chargés de recherche recrutés avant 2021 bénéficieront également de ces nouvelles mesures, grâce à un effort supplémentaire de 26 millions d'euros. Au-delà, ce qui nous disqualifie bien souvent dans la course internationale aux talents, c'est le peu de moyens qu'on donne à nos jeunes chercheurs pour démarrer leurs travaux. Pour éviter de tuer dans l'oeuf leurs premiers élans, ils pourront désormais, grâce à la programmation, compter sur un accompagnement de 10 000 euros en moyenne pour se lancer. lancer. Ce sont bien tous nos personnels de recherche qui feront l'objet du plus grand plan de revalorisation salariale depuis des décennies. Chaque année jusqu'en 2027, 92 millions d'euros supplémentaires y seront consacrés par tranches cumulatives, ce qui représentera un effort global de 2,5 milliards d'euros. Cette enveloppe budgétaire permettra d'harmoniser par le haut les régimes indemnitaires au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche, avant d'engager une convergence interministérielle, afin que nos personnels scientifiques soient traités avec la même considération que les autres agents de l'État à l'horizon 2030. Ces dispositions ont été construites en concertation étroite avec les syndicats. À cet égard, je rappelle que la présente programmation a été examinée par dix-sept instances consultatives.

Ce protocole concerne toutes les fonctions, tous les corps, tous les grades. Par-delà son abord technique, il reconnaît la science comme une oeuvre collective à laquelle chacun apporte sa pierre : celui qui publie les résultats d'une expérience comme celui qui a réglé les instruments, celui qui dirige un laboratoire comme celui qui en assure la logistique, celui qui transmet la connaissance en amphi comme celui qui la valorise dans l'innovation. La reconnaissance du collectif de recherche se traduit par des améliorations très concrètes et très rapides dès 2021, les maîtres de conférences gagneront près de 1 000 euros de plus, les chargés de recherche près de 1 300 euros. Trois plans massifs de repyramidage seront mis en oeuvre au bénéfice des maîtres de conférences, pour porter de 15 000 à 18 000 le nombre de professeurs des universités

Par ailleurs, ce protocole ouvre davantage l'accès aux postes de professeur des universités, aujourd'hui hors de portée de la majorité de nos maîtres de conférences. Au cours des dix prochaines années, 1 500 maîtres de conférences hors classe et 500 maîtres de conférences de classe normale pourront accéder au corps des professeurs. Un horizon bouché a pu conduire certains d'entre eux à chercher d'autres opportunités à l'étranger, ce qui représente un risque majeur pour notre système d'enseignement supérieur et de recherche, qui repose en grande partie sur leur dévouement. C'est dans ce même souci d'attractivité que ce projet de loi crée un nouvel outil : les chaires de professeur junior. Ce dispositif a fait couler beaucoup d'encre et cristallisé bien des inquiétudes. Aussi me permettrez-vous de revenir sur la réalité de son mécanisme : il s'agit de recruter un scientifique sur contrat, après un examen par une commission indépendante, et de l'intégrer dans le corps des professeurs d'université ou des directeurs de recherche au bout de six ans, si l'évaluation finale est positive. Autrement dit, c'est une voie supplémentaire de recrutement. Ni plus ni moins. Elle n'a pas vocation à se substituer au parcours académique classique ni à réduire les perspectives des uns pour améliorer celles des autres. En revanche, elle a vocation à ouvrir le champ des possibles pour tous les établissements trouveront là un levier de plus pour attirer des talents très disputés sur le plan international et aujourd'hui captés par nos voisins sur des dispositifs d'accueil similaires. Les chercheurs désireux de venir ou de revenir en France après un début de carrière à l'étranger trouveront là un moyen de poursuivre leur parcours dans notre pays sans tout reprendre à zéro. nos maîtres de conférences et nos chargés de recherche, ce sont des opportunités nouvelles pour avancer dans leur propre carrière, car chaque recrutement pour une chaire de professeur junior sera accompagné d'au moins une promotion dans le corps des professeurs des universités ou des directeurs de recherche. Ce dispositif est donc bien loin d'être un cheval de Troie destiné à mettre à bas le statut, comme certains le prétendent. C'est au contraire un tremplin pour rendre plus accessibles les carrières académiques, au bénéfice de ceux qui en sont évincés ou qui partent très tôt à l'étranger. Bien au contraire, le niveau de recrutement des enseignants-chercheurs et des chercheurs sera garanti. L'emploi titulaire sera renforcé par la création de 5 200 postes supplémentaires, tout particulièrement dans le champ du soutien à la recherche. C'est tout un pan de l'emploi scientifique que nous avons laissé s'éroder durant la dernière décennie, au point que nos laboratoires souffrent aujourd'hui d'une véritable pénurie d'ingénieurs et de techniciens. Leur savoir-faire est un ingrédient essentiel à la réussite des projets de recherche, que nous n'avons pas su reconnaître ni préserver à sa juste valeur. C'est pour sortir de ce déni qu'il nous fallait aussi apporter une solution concrète à la situation ubuesque dans laquelle se trouvent aujourd'hui les ingénieurs et techniciens non titulaires. Recrutés spécifiquement pour accompagner un projet de recherche sur financements propres, ils en voient rarement l'aboutissement, car leur laboratoire est bien souvent contraint de se séparer d'eux en cours de route, faute de pouvoir renouveler leur CDD. Autrement dit, les outils de recrutement dont disposent actuellement nos laboratoires sont déconnectés de la réalité scientifique. La création du CDI de mission scientifique vient résoudre ce hiatus, en permettant à la durée du contrat d'épouser la durée du projet. Derrière cette rationalisation des procédures et cette synchronisation du temps scientifique et du temps administratif, il y a aussi un indéniable progrès social pour des milliers d'agents non titulaires là où notre système les condamne aujourd'hui à la course incessante aux CDD, ce nouvel outil leur offrira la protection, les garanties et les droits afférents au CDI. Pour nos laboratoires, c'est autant de temps et d'énergie en plus pour la recherche. En ce sens, la création du CDI de mission scientifique participe du troisième axe de ce projet de loi, à savoir la simplification de la vie des laboratoires. Cet aspect de la programmation est pour moi essentiel. Le quotidien de la recherche constitue en effet l'angle mort des réformes structurelles de ces dernières décennies. Pendant que l'on démontait et remontait le meccano institutionnel, nous n'avons pas vu que les procédures, les formulaires, les dossiers d'évaluation, les demandes de financement se démultipliaient, envahissant la vie des laboratoires jusqu'à l'asphyxie. À ceux-ci, il est grand temps de redonner du souffle, comme il est grand temps de rendre les chercheurs à la recherche. Mais pour y parvenir, il faut se donner la peine d'enfiler la blouse et de penser à hauteur de paillasse ; c'est pourquoi il était si essentiel d'associer de très près la communauté à l'élaboration de ce texte. C'est grâce à ce regard de terrain, qui est aussi le mien, que nous proposons aujourd'hui une série de mesures concrètes dont l'abord parfois trivial ne doit pas masquer l'impact majeur sur le quotidien de nos chercheurs. Supprimer l'autorisation administrative préalable au cumul d'activités, référencer l'ensemble des appels à projets sous un portail unique, harmoniser les calendriers et les cahiers des charges sont autant de petites victoires contre la machine administrative et de précieuses heures rendues chaque jour à la science. D'autres simplifications verront le jour dans le cadre du vaste chantier de simplification ouvert par cette programmation. telles respirations doivent être introduites aussi dans la carrière des enseignants-chercheurs, qui voient trop souvent leur charge d'enseignement prendre le pas sur le temps dévolu à leurs travaux de recherche. Afin de les aider à trouver un meilleur équilibre entre leurs deux missions, la programmation élargit l'accès aux congés pour recherches ou conversions thématiques, aux délégations du CNRS ainsi qu'à l'Institut universitaire de France, autant de dispositifs qui offrent aux enseignants-chercheurs la possibilité de se consacrer plus librement à leurs recherches durant une période dédiée. Mesdames, messieurs les sénateurs, tout ce temps, cette visibilité, ces moyens rendus à la recherche par le biais de cette programmation, c'est, en réalité, autant de temps, de visibilité et de moyens rendus à notre pays pour aborder les prochaines décennies avec confiance. Investir dans la recherche, c'est investir dans notre avenir commun. C'est pourquoi il est si essentiel de remettre la recherche au coeur de la vie économique et culturelle de notre pays. Telle est la clé de voûte du texte que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. J'ai évoqué, au début de cette intervention, le décalage entre l'excellence de nos formations et la fuite de nos cerveaux. En réalité, là n'est pas le seul paradoxe de la science française : nous devons aussi nous interroger sur le hiatus entre l'excellence de notre recherche académique et la faiblesse de ses retombées économiques. À l'heure de la relance, alors que l'ombre de la crise plane sur leur compétitivité, nos start-up, nos PME, nos entreprises ont plus que jamais besoin de puiser dans nos laboratoires le surcroît d'innovation qui fera la différence dans la compétition internationale. Le potentiel est énorme : parmi les 83 start-up qui ont récemment rejoint le programme French Tech 120, qui identifie les pépites les plus susceptibles de devenir des leaders technologiques de rang mondial, 17 sont issues de la recherche publique- et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Pour réaliser toutes les promesses de la recherche académique, il nous faut résolument accélérer le transfert des connaissances entre nos laboratoires et nos entreprises. Or cette programmation, qui prend à bras-le-corps le défi de l'attractivité des carrières scientifiques en France, se saisit avec le même pragmatisme ambitieux des enjeux d'innovation. Tant les hommes que les idées doivent circuler d'un monde à l'autre. C'est pourquoi la programmation prévoit, d'une part, de favoriser les mobilités public-privé, en autorisant les chercheurs à consacrer plus de temps à la création de leur start-up ou à la vie d'une entreprise, et en facilitant la démarche des doctorants désireux d'effectuer leur thèse dans le privé, grâce à l'augmentation de 50 % du nombre de bourses Cifre, et à la définition d'un contrat doctoral de droit privé. Et c'est pourquoi elle prévoit, d'autre part, de stimuler la recherche partenariale en doublant les financements de l'ANR consacrés aux chaires industrielles, aux laboratoires communs et aux instituts Carnot, et en labellisant les sites universitaires qui auront su rendre leur offre de transfert plus simple, plus lisible et plus rapide. rapide. S'il est un autre dialogue qui doit gagner en intensité et en familiarité, c'est celui de la science et de la société. La crise que nous traversons jette une lumière crue sur leurs relations ambiguës : certains de nos concitoyens s'irritent de la démarche tâtonnante de la science et de ses controverses, d'autres caricaturent ses valeurs en confondant doute méthodique et complotisme ; mais, en définitive, tous attendent d'elle des repères dans le brouillard et scrutent l'horizon de la recherche dans l'espoir de voir poindre un traitement et un vaccin. Car, en vérité, à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective, nous avons besoin de science dans nos vies, pour rendre celles-ci moins opaques et moins incontrôlables, pour les rendre plus dignes d'être vécues, pour les rendre moins solitaires, parce que la démarche scientifique et son esprit de raison nous ouvrent aussi la voie du débat et de l'altérité. La science a ceci de commun avec l'art qu'elle permet de vivre un ton plus haut, et personne ne peut ni ne doit être privé de cette dimension supérieure. Cette programmation porte donc l'ambition de ménager une vraie place à la recherche dans les esprits, dans les foyers et dans l'espace public en encourageant les scientifiques à aller au-devant de la société, et la société à revendiquer sa place auprès des scientifiques. Il s'agit bien d'instaurer un véritable partage de la science, d'une part, en stimulant les recherches participatives, et, d'autre part, en soutenant les chercheurs qui s'impliquent dans la médiation scientifique, auprès du grand public, auprès des jeunes, auprès des médias, notamment au travers d'initiatives comme « Une classe, un chercheur » ou grâce à des lieux innovants permettant des échanges entre journalistes et scientifiques. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, vous l'aurez compris, le projet que je porte devant vous, c'est la possibilité d'un chemin pour notre recherche. Programmer la recherche, c'est construire dès à présent l'édifice qui résistera aux aléas de l'avenir. Ce n'est pas seulement faire un pari sur la connaissance, c'est faire le choix de la connaissance

Bien sûr, voir le monde à travers les yeux du savoir est exigeant ; c'est parfois même inconfortable, car il faut accepter de vivre avec une part d'incertitude et une part d'irrésolution. Telle est pourtant la seule démarche qui nous garantit de faire des choix responsables et engagés, d'agir en hommes et en femmes libres, en cultivant, au sens le plus concret de ce terme, le rêve d'un monde meilleur. C'est pourquoi la science est la meilleure alliée de la démocratie, de la décision politique, du débat citoyen, et c'est pourquoi je sais pouvoir compter sur tout votre engagement dans les discussions qui s'ouvrent aujourd'hui autour de ce texte majeur pour l'avenir de notre pays. La parole

c'est pour moi un grand honneur d'ouvrir cette discussion au Sénat sur le projet de loi de programmation de la recherche. Au milieu des tumultes d'une actualité quotidienne peu réjouissante, il est essentiel pour nous tous de continuer à construire, brique par brique, le futur de nos enfants et de notre pays. perspective, le sujet de la recherche est structurant. Nous le savons, en effet : nous sommes entrés, sans y être toujours bien préparés, dans une ère où la puissance d'une nation ne se mesure plus à sa capacité à produire, mais à sa et donc à miser sur les techniques innovantes dans tous les domaines : systèmes numérisés, nanotechnologies, nouvelles énergies, biologie, santé. Programmer le financement et le fonctionnement de la recherche, valoriser le statut de celles et ceux qui s'y consacrent, c'est donc tracer la route de notre destin collectif. Le projet de loi que nous allons examiner n'est pas un document de plus, perdu dans l'abondante production législative de notre pays. Ce texte devrait servir de ligne d'horizon à la plupart de nos décisions. Il dépasse les enjeux d'opinion et les postures. Nous allons en débattre sans jamais perdre de vue qu'il doit dessiner notre avenir partagé. La commission, dans des conditions rendues difficiles par la proximité du renouvellement sénatorial, sans même évoquer la modification de l'ordre du jour dont nous avons été informés hier, a mené un travail approfondi et serein. Je veux ici saluer mes collègues de tous les groupes qui ont participé aux très nombreuses auditions que nous avons menées. Un premier élément nous a, me semble-t-il, tous frappés : c'est l'attente très forte parmi la communauté des chercheurs non seulement de moyens budgétaires- nous allons y revenir mais aussi, et surtout, d'une vraie reconnaissance de leur rôle éminent dans notre société fragilisée par l'épidémie de covid-19 et fracturée par les fausses informations. Nous devons en avoir conscience, mes chers collègues : de très nombreux chercheurs auront aujourd'hui les yeux braqués sur cet hémicycle et attendent un débat à la hauteur des enjeux. Ce débat, nous le leur devons. Dès lors, posons-nous la question de manière « scientifique » les promesses portées par ce texte sont-elles tenues ? Je vais hélas ! devoir apporter une réponse mesurée et nuancée, tout d'abord, parce que les attentes étaient à la hauteur de la situation très difficile dans laquelle doit vivre, parfois survivre, notre recherche. Je veux rappeler quelques données : avec un niveau de financement de la recherche publique et privée qui stagne autour de 2,2 % du PIB depuis plus de vingt la France a accumulé un retard excessif, abandonnant à d'autres pays européens le leadership en matière de recherche et d'innovation. Illustration terrible de cette situation pour notre fierté nationale- vous l'avez évoquée, madame la ministre -, Emmanuelle Charpentier, jeune prix Nobel de chimie cette année, a expliqué qu'elle n'aurait jamais pu mener ses recherches pionnières et majeures en France. Ce cas ne relève pas de la simple anecdote : quand un chercheur de ce niveau fait le choix de poursuivre ses recherches à l'étranger, il emporte avec lui son aura, ses financements, ses compétences ; il ne fera pas bénéficier les jeunes chercheurs français de ses connaissances. La facture du manque d'engagement de ces dernières années, c'est maintenant que nous la payons. Évitons à nos enfants de vivre, dans vingt ans, dans un pays déclassé, alors même que tout concourt à notre excellence. Je veux mettre à votre crédit, madame la ministre, votre grande connaissance du milieu de la recherche et de l'enseignement supérieur, dont vous êtes issue, ainsi que votre volontarisme, qui a permis, dans un contexte où tout invite à se concentrer sur l'urgence, d'inscrire à l'ordre du jour un projet de loi préparant justement l'avenir. C'était nécessaire et courageux. ? Quelle est son ambition ? Si nous devions porter une appréciation sur la copie, nous serions nombreux, me semble-t-il, à écrire : « Peut mieux faire ». Car le meilleur baromètre de l'attention que porte une nation à sa recherche, ce sont les moyens De ce point de vue, et même si nous aurons un débat technique à l'article 2, convenons que la durée de la programmation, jamais vue sous la V République, démontre moins un engagement au long cours qu'une volonté de décaler les échéances budgétaires Sur la période de dix ans que vous proposez, l'effort est en réalité bien plus limité que celui qui est affiché, si l'on tient compte de l'inflation. Certes, on pourrait à raison objecter qu'un engagement de plus de 25 milliards d'euros en cumulé constitue déjà un changement de cap majeur par rapport au sous-investissement chronique que la recherche subit depuis plusieurs décennies. Cependant- nous le savons -, une loi de programmation de cette durée, c'est hélas ! plus du sable que du marbre. Je résume : crédits insuffisants pour rattraper notre retard, d'une part, faible garantie sur leur réelle disponibilité, d'autre part. Comment susciter la confiance à grande échelle dont nous avons besoin et que la communauté appelle de ses voeux ? Je ne doute pas, madame la ministre, de votre mobilisation ; j'imagine que les débats internes au sein d'un gouvernement peinant à établir ses priorités ont dû être intenses et que, peut-être, l'accord obtenu sur la loi de programmation examinée à partir d'aujourd'hui constitue un point d'équilibre ... Permettez-nous cependant de trouver cet équilibre encore insatisfaisant. La commission de la culture, de l'éducation et de la communication a cherché à donner un peu plus d'ampleur à votre texte, suivant quatre axes. Le premier axe, que nous avons proposé conjointement avec les commissions des finances et des affaires économiques, consiste à ramener, à enveloppe constante, la durée de la programmation à sept ans. Pourquoi sept ans ? Parce que cette durée, plus conforme à celle qui est habituellement choisie pour les lois de programmation, permet de limiter les conséquences des aléas politiques et économiques sur la trajectoire initiale, d'aligner la recherche française sur le calendrier du programme-cadre européen et d'accroître l'intensité de chaque marche budgétaire annuelle, un effort particulier étant consenti les deux premières années. C'est bien une trajectoire plus crédible, plus rapide et plus efficace que nous proposons pour provoquer le sursaut budgétaire dont notre recherche a besoin. Deuxième axe : offrir des garanties aux chercheurs et veiller à la place des femmes. La commission a globalement accueilli avec intérêt les nouveaux dispositifs de recrutement contenus dans le projet de loi. Elle a cependant tenu à apporter des garanties à leurs bénéficiaires, en instaurant une durée minimale pour le contrat de mission scientifique, en veillant à ne pas allonger de manière excessive le contrat postdoctoral, et en prévoyant la possibilité de prolonger les contrats doctoraux et postdoctoraux en cas de congé maternité, de congé paternité, de congé maladie ou de congé pour accident du travail. Concernant les chaires de professeur junior, qui suscitent des inquiétudes légitimes au sein de la communauté scientifique, la commission a abaissé à 15 % le pourcentage limite de recrutement annuel autorisé afin de mieux traduire le caractère très spécifique de ce dispositif, qui n'a pas vocation à se substituer aux voies de recrutement traditionnelles. La commission a aussi souhaité valoriser, dans la carrière des chercheurs et enseignants-chercheurs, les actions que ceux-ci mènent en direction des citoyens pour favoriser la diffusion des connaissances. ailleurs soulevé la question des inégalités entre les femmes et les hommes dans l'accès à certaines disciplines, à certaines responsabilités et à certaines formes de financement. Si la traduction de cette préoccupation en mesures législatives, et non seulement déclaratives, est parfois malaisée, la commission est convaincue que l'égalité entre les femmes et les hommes doit constituer, pour le monde de la recherche, une priorité structurante dans les prochaines années. Troisième axe, dont nous aurons à débattre dans cet hémicycle : l'affirmation de l'intégrité scientifique et des libertés académiques dans la loi. Ces deux sujets, distincts mais intimement liés, ont donné lieu à un travail transpartisan qui, je le crois, honore notre assemblée et montre notre capacité à élever nos convictions au niveau des enjeux. Ne nous y trompons pas : intégrité scientifique et libertés académiques ne sont pas, pour les chercheurs, de vains mots. Elles définissent rigoureusement un espace de liberté, mais également de principes à suivre. La position à laquelle nous sommes parvenus ne répond pas seulement à l'actualité, même si cette dernière, tragique, est présente à nos esprits. Elle vise bel et bien à bâtir un corpus de droits et de devoirs qui fonde l'exercice professionnel des chercheurs et des enseignants-chercheurs. Quatrième axe structurant pour notre travail : la nécessaire implication des collectivités territoriales, grandes absentes du texte initial. Pour pallier ce manque regrettable, la commission a ajouté un volet territorial aux contrats de site conclus entre l'État et les établissements partenaires d'un même site universitaire. Vous l'avez compris : nous avons, sur ce projet de loi, réellement travaillé au plus près des préoccupations très nombreuses dont nous avons été saisis. Ce que nous regrettons, au fond, c'est le défaut d'ampleur de ce texte, qui aurait pu et dû porter des moyens et une vision plus affirmés pour les prochaines années. De cette ambition limitée et de ce débat que nous avons dans des conditions si étranges, il ressort l'impression d'une forme d'inachevé. Je vais cependant m'efforcer de demeurer résolument optimiste comme je le disais dès mes premiers mots, malgré son aspect technique, parfois aride, et en dépit de la diversité des propositions qu'il contient, touchant notamment à la simplification des procédures, de loi est un, une ligne de conduite pour notre pays, qui doit rester compétitif dans un secteur qui conditionne tous les autres : celui de la recherche et de l'innovation, lesquelles relèvent toutes deux de la longue durée. Il n'est guère d'autre domaine qui nécessite à ce point une vision programmatique. J'espère que nos travaux nous aideront à affronter les défis du futur. C'est là l'essentiel. Et c'est ce que la Nation attend de nous. Merci, madame la rapporteure,

la commission des affaires économiques a d'abord regretté que ce projet de loi, et en particulier la trajectoire budgétaire qui y est présentée, soit centré sur la recherche publique rattachée au ministère de la recherche. que c'est par facilité -de ne faire porter ce projet de loi que par un seul ministère, le Gouvernement a, me semble-t-il, manqué ici une occasion de lancer un grand chantier pour en finir avec le morcellement des politiques de recherche et développement et d'innovation. J'en viens directement à ce que contient ce projet de loi. Je ne rappellerai pas ce que nous savons tous déjà, à savoir que la situation de la recherche française est grave et mérite d'être redressée par le biais de moyens qui soient à la hauteur de nos ambitions. Pour cette raison, la commission des affaires économiques a voté,

Madame la ministre, puisqu'il s'agit de redonner des moyens aux opérateurs de recherche, je me permets d'insister sur un point que nous avions déjà évoqué lors de votre audition par la commission de la culture les opérateurs de recherche sont contraints d'appliquer une norme comptable inadaptée, qui les oblige à garder en trésorerie des centaines de millions d'euros ! C'est autant d'argent qui n'est pas fléché vers les laboratoires. Il faut faire évoluer les choses, et il faut, si vous le pouvez, le faire rapidement Ce projet de loi traite par ailleurs d'une thématique importante pour la commission des affaires économiques, à savoir le resserrement des liens entre la recherche publique et les entreprises ; c'est opportun. Concernant la réintroduction du dispositif de congé d'enseignement ou de recherche, dont le principe est assurément bienvenu, notre commission a estimé qu'il fallait laisser plus de place à la négociation collective et éviter de faire peser des charges excessives sur les petites entreprises, compte tenu du contexte. Sur ce sujet des liens avec les entreprises, je me permettrai une remarque : le Gouvernement envoie deux messages contradictoires. D'un côté, avec ce texte, on souhaite inciter les laboratoires à développer des relations avec les entreprises. De l'autre, avec le projet on ôte le principal outil d'incitation des entreprises à se tourner vers la recherche publique, à savoir le doublement de l'assiette du crédit d'impôt recherche en cas de recours à un laboratoire public. Cette mesure risque d'anéantir les efforts du Gouvernement en la matière. Je sais que l'on ne peut pas faire autrement, car une plainte, que nous aimerions, d'ailleurs, pouvoir consulter, a été déposée auprès de la Commission européenne. Mais si nous n'avons vraiment pas le choix, il faut,, prévoir des compensations. Madame la ministre, toute la communauté est inquiète à ce sujet J'en viens maintenant aux ordonnances portant sur des secteurs relevant des compétences de notre commission, à savoir l'agriculture et le spatial. Nous avons retenu une ligne de conduite là où les marges de manoeuvre du législateur sont limitées par des textes ou des jurisprudences, et dans la mesure où il s'agit de sujets techniques, nous n'avons rien trouvé à y redire. En revanche, lorsqu'il s'agit de sujets importants, dont nous estimons qu'ils méritent un vrai débat parlementaire, nous avons proposé la suppression des habilitations à légiférer par ordonnance. C'est le cas pour deux de ces habilitations, qui donnent de véritables blancs-seings au Gouvernement. Il s'agit des ordonnances relatives, d'une part, à la redéfinition des procédures d'édiction d'avis relatifs aux biotechnologies, et, d'autre part, à la refonte de la loi relative aux En conclusion, la commission des affaires économiques considère que ce projet de loi va dans le bon sens, mais qu'il mérite d'être musclé, ce qui a été fait par nos trois commissions. Je souhaite d'ailleurs remercier de nouveau Mme la rapporteure de la commission de la culture de son écoute et de la qualité de son travail, ainsi que M. le rapporteur pour avis de la commission des finances de l'éclairage financier qu'il a su donner sur ce texte.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après avoir repoussé à plusieurs reprises sa présentation, le Gouvernement a finalement déposé le 22 juillet dernier un projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030. Vous l'avez rappelé, madame la ministre : il s'agit de donner de la visibilité aux acteurs de la recherche, en dessinant une trajectoire à même de porter nos dépenses de recherche à 3 % du PIB à l'horizon 2030. notre pays est confronté à un risque bien réel de décrochage par rapport aux autres pays qui sont à la pointe de la recherche. Tandis que nos principaux concurrents consacrent une part croissante de leur richesse nationale à cet effort, nos dépenses publiques de recherche stagnent depuis une dizaine d'années, avec une croissance en volume de l'ordre de 1,3 % entre 2008 et 2018. La dépense de recherche des administrations a même reculé de 2,2 % entre 2015 et 2018 Faisons-nous encore partie des grands pays de la recherche ? Il me semble que oui. Pourrons-nous en dire de même dans dix ans ? Si nous ne nous décidons pas à inverser la tendance et à investir massivement dès aujourd'hui dans notre recherche, rien n'est moins sûr. Vous l'avez compris, madame la ministre : un sursaut est nécessaire ; tel est l'objet du présent texte. J'en partage, dans les grandes lignes, les orientations. Il s'agit, en premier lieu, de revaloriser les métiers de la recherche, pour attirer les plus grands talents, mais surtout pour retenir nos chercheurs les plus prometteurs. À cet égard, l'exemple récent d'Emmanuelle Charpentier, lauréate française du prix Nobel de chimie 2020 ayant effectué l'intégralité de ses travaux à l'étranger, illustre tristement la fuite des cerveaux à laquelle nous sommes confrontés.

Si le renflouement de l'ANR était donc indispensable, il ne doit pas avoir pour corollaire une attrition des moyens récurrents dont disposent les laboratoires. Il doit également s'accompagner d'une simplification des procédures, afin de faciliter le quotidien de nos chercheurs, qui sont trop souvent confrontés à de véritables parcours du combattant quand ils candidatent auprès des différentes agences. Pour conclure sur les grandes orientations de ce texte, je regrette que certains pans de la politique de recherche soient passés sous silence. Je pense notamment au devenir du crédit d'impôt recherche, à l'articulation avec les échelons infranationaux et supranationaux, ou encore à la participation française aux appels à projets européens. J'en viens maintenant à la programmation budgétaire. Si je partage les grandes orientations définies par le Gouvernement, je suis en revanche nettement plus dubitatif quant à la traduction budgétaire de ces orientations. En effet, sur le papier, si j'ose dire, la trajectoire pourrait à première vue paraître satisfaisante. Mais, en réalité, madame la ministre, certains de vos choix programmatiques jettent un doute sérieux sur la crédibilité et la sincérité de cette trajectoire. Tout à fait. En premier lieu, j'attire votre attention sur le fait que la programmation ne tient pas compte des effets de l'inflation.

Je tiens donc à lever toute ambiguïté : en cumulé sur la période 2021-2030, la recherche publique ne bénéficiera pas de 25 milliards d'euros, mais de 7,2 milliards d'euros supplémentaires, c'est-à-dire un quart de l'effort annoncé Je suis bien conscient de l'imprévisibilité qui caractérise la conjoncture économique actuelle ; cependant, j'estime que les projections réalisées mettent en lumière le caractère très incertain de la trajectoire que vous nous présentez aujourd'hui. De toute évidence, madame la ministre, il vous faut admettre que cette trajectoire ne permettra pas de porter les dépenses de recherche des administrations à 1 % du PIB- c'est impossible. En réalité, elle se bornera à stabiliser la part des dépenses de recherche dans le PIB. Dans ce contexte et à la lumière de ces éléments, le choix d'une programmation sur dix ans me paraît particulièrement inapproprié, car nuisant à la crédibilité de la trajectoire. Qui plus est, ce choix se traduit par des marches annuelles trop faibles pour provoquer le sursaut dont notre pays a besoin.

Madame la ministre, je suis conscient des contraintes budgétaires actuelles. J'estime néanmoins que les deux premières années de la programmation seront essentielles pour notre recherche, et qu'il faut à tout prix prévoir une accélération considérable de cette trajectoire. Dans ce contexte, je serais favorable à ce qu'une part supplémentaire des crédits dédiés à la relance vienne abonder la loi de programmation. conclure, une phrase de Marie Curie : « Rien n'est à craindre, tout est à comprendre. » Je ne crains pas votre loi de programmation de la recherche, madame la ministre ; j'aimerais simplement en comprendre les tenants et les aboutissants financiers. Je suis saisi,

en 2030. Et nombre de nos collègues dénoncent à raison des effets d'annonces dépourvus de toute prise avec la réalité de la recherche et de l'enseignement supérieur. La chambre haute, réputée pour sa sagesse, préconise d'ailleurs quasi unanimement de ramener la durée d'engagement de dix à sept ans, d'une part, parce que cela serait plus conforme aux autres programmations, d'autre part, parce qu'il y a, là encore, une forme de malhonnêteté intellectuelle à faire supporter par les majorités à venir l'essentiel de l'effort budgétaire, tout particulièrement dans le contexte que nous connaissons actuellement. Au contraire, parce que les retards pris confinent au décrochage, il est nécessaire d'enclencher dès maintenant une trajectoire volontariste et ambitieuse, un « choc », comme on dit maintenant, pour que les investissements de la France dans sa politique de recherche Car le désengagement a des conséquences bien réelles sur le quotidien de celles et ceux qui font vivre la recherche dans notre pays, mais aussi sur les capacités de notre pays et de notre société à se hisser au niveau des enjeux de notre époque. Depuis des années, les chercheurs alertent sur les initiatives nationales et internationales auxquelles ils doivent renoncer, malgré l'intérêt et l'apport scientifiques de celles-ci. Ils alertent sur le sous-financement chronique de leurs travaux

Comment comprendre que David Veesler ait finalement fait le choix de partir pour Washington afin de poursuivre ses travaux sur les maladies infectieuses et les coronavirus ? Mes chers collègues, les chercheurs l'ont dit durant les auditions, à l'instar de Christophe d'Enfert : ils manquent de moyens et de visibilité, et sont contraints de se disperser dans des procédures longues et peu productives pour obtenir des financements souvent insuffisants. C'est à cette réalité que ne s'attaque pas cette loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR). À cet égard, le projet de loi de finances pour 2021, également examiné en ce moment même, montre la fragilité des promesses financières. Ainsi, les dépenses d'investissement devraient baisser cette année de près de 17 %. Quant à la désignation

de la recherche spatiale ou encore de l'intégration des licences professionnelles dans Parcoursup, autant de sujets qui suscitent objectivement le débat. Un débat qu'il faut mener démocratiquement et au grand jour. Dans le contexte sanitaire actuel, à quelques heures de nouvelles annonces qui impacteront profondément la vie sociale de nos concitoyens, l'économie de la France et même notre démocratie, le rôle de la recherche n'aura jamais été aussi crucial. Je pense bien entendu à la recherche publique, pour laquelle l'État n'assume pas son rôle. Le projet de loi de finances en discussion à l'Assemblée nationale est édifiant de ce point de vue. En pleine crise sanitaire, alors même que les enjeux de transition écologique sont si forts, la recherche en santé

les travaux lancés par cette équipe sur les coronavirus sont-ils bloqués par l'absence d'un cryo-microscope électronique ? Le microscope dont ils disposent actuellement n'est pas adapté à la nature des recherches en cours, faute d'une résolution suffisante. Oui, la période que nous traversons nécessite un traitement de choc en matière de recherche. C'est également vrai en matière de recherche privée. Reconquérir une industrie digne de ce nom en France, relocaliser des productions, retrouver notre souveraineté dans des domaines stratégiques, cela implique d'impulser, voire de se contraindre à un plus grand effort aussi en matière de recherche privée. Comment accepter, par exemple, que telle industrie pétrochimique abandonne une unité de recherche travaillant sur le caoutchouc, laquelle était en mesure d'inventer les matériaux de demain permettant d'alléger le poids des véhicules, quand, parallèlement, la puissance publique décide de pénaliser financièrement les modèles les plus lourds afin de diminuer la pollution ? Comment se résigner au plan social en cours chez Boiron, que la direction du groupe justifie par le déremboursement progressif de l'homéopathie, alors qu'il y aurait besoin de rapatrier des productions pharmaceutiques dans notre pays ? Chacun de ces exemples- on pourrait en citer d'autres -montre que les renoncements du secteur privé en matière de recherche sont en cause. Ces renoncements sont d'autant plus importants que la puissance publique délaisse elle-même son propre rôle. Une nouvelle fois, la question du crédit d'impôt recherche est posée, et vous ne serez pas surpris que nous y revenions. Sans chercheurs, il n'y a pas de recherche. À ce titre, la baisse constante du nombre de doctorants ne peut que nous inquiéter. De la même manière, l'appui administratif fait aujourd'hui fortement défaut aux équipes de recherche, notamment dans le cadre des recherches de financement. Là encore, le projet 2021 prévoit une baisse des dépenses de personnel de plus de 12 %. Le Conseil d'État et le Conseil économique, social et environnemental (CESE) ont parfaitement illustré la chose. En multipliant la création des contrats précaires, de chaires de professeur junior en CDI de mission, en passant par le contrat doctoral privé, vous optez pour une recherche de court terme et non pour des programmes ambitieux. ignorez totalement, au passage, la Cour des comptes, qui pointait la surreprésentation des contractuels au sein de votre ministère. En matière de personnels, vous avez renvoyé aux universités, et ce à plusieurs reprises, la responsabilité des postes non pourvus, malgré des plafonds d'emplois relevés depuis 2018. C'est oublier un peu vite que, si les universités utilisent allègrement le mécanisme de « fongibilité asymétrique c'est pour faire face au sous-financement chronique des établissements et compenser, notamment, le renoncement de l'État à financer le glissement vieillesse technicité Et que dire de la rémunération de nos chercheurs, moins payés que chez nos voisins ? Un protocole d'accord sur les rémunérations et les carrières vient d'être signé, mais les crédits qui devraient permettre sa concrétisation ne sont inscrits nulle part mon propos sur le fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche. Cette dernière, malmenée par des baisses récurrentes de crédits, reste encore largement contre-productive. Malgré votre volonté d'en améliorer le fonctionnement, nous doutons que l'outil soit véritablement pertinent. En effet, cette agence participe pleinement à l'écosystème de l'enseignement supérieur concurrentiel et tourné vers le classement de Shanghai. Or, comme on le voit avec les initiatives d'excellence (IDEX) et le programme d'investissements d'avenir (PIA), notamment, cette stratégie de pôles d'excellence dévoie le modèle de service public national d'enseignement supérieur. Je m'inquiète à ce titre de la moyen terme, des universités de taille plus réduite. On constate d'ores et déjà la concentration des financements d'avenir dans les métropoles et de grandes inégalités de financement entre domaines d'études, au détriment notamment des sciences humaines et sociales. Pourtant, c'est bien ce modèle concurrentiel que le projet de loi alimente et poursuit. Beaucoup d'entre vous en êtes conscients, mes chers collègues, comme en témoignent les nombreuses réactions sur la nécessité de prendre en compte les enjeux d'aménagement du territoire, eux aussi trop absents de ce Ce texte suscite, depuis sa parution, de nombreuses oppositions de la part d'enseignants, de chercheurs, de maîtres de conférences. Vous l'avez sûrement constaté, mes chers collègues, au vu de la vague de méls que vous avez reçus. Adoption de motions lors d'assemblées générales d'unités de recherche ou du Comité national de la recherche scientifique, 814 directeurs de laboratoire prêts à démissionner de leurs responsabilités administratives, avis plus que réservé du CESE, du Conseil d'État, du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE), je n'en jette pas davantage. Écoutons les premiers concernés par ce texte : ils nous disent, unanimement, leur profond désaccord quant à l'avenir proposé pour notre recherche. Par cette motion, nous vous proposons de suivre l'avis de tous les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche,

entre l'innovation et la prospérité. Les nations qui ont dominé leur temps et leur monde ont presque toujours été celles qui ont maîtrisé la modernité, la technicité. « Celui qui voit loin va loin », dit un vieux dicton picard. Aussi, nous le savons tous, la recherche doit être une priorité. Elle l'est souvent dans les discours, elle doit le devenir dans les actes.

dénonce une « profonde inadéquation entre les ambitions nécessaires et l'insincérité manifeste du contenu de la loi de programmation ». Les travaux de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, saisie au fond, ainsi que des deux commissions, celles des affaires économiques et des finances, saisies pour avis, ont effectivement pointé un effort budgétaire insuffisant et une trajectoire peu crédible de ce projet de loi, malgré les effets d'annonce du Gouvernement. La trajectoire budgétaire prévue initialement s'étendait sur dix ans pour atteindre, à terme, un supplément annuel de 5 milliards d'euros,

-a établi qu'en euros constants, c'est-à-dire une fois neutralisés les effets de l'inflation, la hausse prévue à l'horizon 2030 par la loi de programmation serait environ quatre à cinq fois inférieure à ce qui était annoncé. Cela revenait seulement à stabiliser la part des dépenses de recherche dans le PIB. ailleurs, il n'y a jamais eu précédemment de trajectoire fixée sur dix ans. Cette durée inhabituellement longue, comme l'a souligné le Conseil d'État, l'exposait à des aléas aussi bien politiques qu'économiques, et faisait reposer la plus grande part de l'effort budgétaire sur l'après-quinquennat.

l'effort budgétaire proposé ne pouvait permettre d'atteindre l'objectif de Lisbonne de 1 % du PIB en faveur de la recherche publique, ce qui a été confirmé par les projections des plus grandes instances scientifiques de ce pays. Notre groupe partage donc le constat figurant dans la motion sur le manque de crédibilité de la programmation proposée par le Gouvernement. Cependant, ce n'est pas ce texte que nous examinons aujourd'hui. La commission de la culture, ainsi que les deux commissions saisies pour avis, ont modifié la trajectoire budgétaire prévue. Elles ont limité sa durée à sept ans et concentré l'effort sur les premières années. Ainsi, elles ont prévu pour 2021 et 2022 des marches successives de 1,1 milliard d'euros à destination des programmes de recherche, soit un abondement de 3,3 milliards d'euros sur deux ans. Le projet initial prévoyait, quant à lui, une hausse moyenne de 450 millions d'euros sur les deux premières années. Ce coup d'accélérateur est indispensable : nous sommes passés en matière de recherche et développement de la quatrième à la douzième place des pays de l'OCDE entre le début des années 1990 et aujourd'hui. Nous ne saurions en être fiers Notre effort public de recherche est passé, dans le même temps, de près de 1 % du PIB à moins de 0,8 %. Or de nombreux pays européens ont déjà atteint l'objectif de Lisbonne. La bataille économique se joue, aujourd'hui plus que jamais, sur le terrain scientifique et technologique. Faire de la recherche l'une des variables d'ajustement budgétaire est un non-sens, et même une faute politique Le texte issu des travaux de nos commissions renoue donc avec l'ambition légitime qu'aurait dû avoir ce projet de loi. Tout d'abord sur le plan financier, comme je viens de l'indiquer, mais également par diverses dispositions visant à améliorer notre système de recherche. Car, si ce texte est dépourvu de grandes mesures structurelles, il aborde des questions concernant directement les chercheurs et les enseignants-chercheurs, telles que leur recrutement, le fonctionnement des organismes de recherche ou les relations avec le secteur privé. Sur chacun de ces thèmes, la commission de la culture, dont la position était très attendue par la communauté scientifique- nous avons en effet tous reçu un nombre impressionnant de méls -, a proposé

La commission s'est attachée à apporter davantage de protection aux doctorants et postdoctorants, afin que les nouveaux contrats créés par le projet de loi soient réellement attractifs- on peut toujours faire mieux, il est vrai ... Elle a amélioré la situation des chercheuses-

afin que nos collectivités puissent être associées aux problématiques de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce sont des enjeux importants, et seule la poursuite de l'examen de ce projet de loi permettra leur concrétisation.

Il s'agit de consolider le texte issu de nos travaux en prévision d'une lecture commune avec les députés. Ainsi, parce que ce projet de loi fixe une trajectoire budgétaire plus ambitieuse et encadre des initiatives favorables audéveloppement de la recherche,

de cette motion relèvent à juste titre les faiblesses du projet de loi : un calendrier d'examen accéléré, une présentation budgétaire difficilement lisible, une trajectoire manquant de sincérité. Cependant, le caractère quelque peu exagéré et sans nuance du constat dressé doit aussi être souligné. L'engagement budgétaire contenu dans ce projet de loi mérite d'être salué, en ce qu'il rompt avec deux décennies de sous-investissement public chronique dans la recherche. Il constitue en cela un changement de cap important. La commission a toutefois décidé de ramener la durée de la programmation à sept ans, au lieu des dix ans retenus par le Gouvernement, pour construire une trajectoire budgétaire plus crédible et plus efficace. Ce faisant, il s'agit d'envoyer un signal fort à la communauté de la recherche, en attendant une véritable ambition pour ce secteur.

qui mobilise la Nation, l'opinion publique et les forces vives du pays. Qu'y a-t-il en effet de plus important aujourd'hui que de préparer l'avenir et de rattraper le niveau d'excellence de la recherche française, qui s'est dégradé depuis des années ? Nous en avons d'autant plus besoin que, dans la période actuelle, le doute scientifique et l'appétence à développer les connaissances et le savoir

de loi prévoit des avancées en termes d'amélioration des carrières, d'attractivité de la recherche, de simplification des mesures et de rénovation des outils de financement.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à la fin des années 1990, le virologue Hubert Laude, seul spécialiste français des coronavirus, internationalement reconnu, a dû se résoudre à arrêter ses recherches, son laboratoire du CHU de Caen fermait, faute d'intérêt et de vision prospective quant aux travaux qu'il menait depuis vingt ans. Outre le caractère amèrement piquant de ce rappel, les conditions des découvertes de l'équipe d'Hubert Laude sont particulièrement instructives. Comme le souligne l'un des membres de son équipe, « tous les résultats ont été obtenus sans financement spécifique, juste avec l'argent de fonctionnement du laboratoire ». Et le virologue de conclure : « La recherche est comme un arbre qui pousse lentement. Il faut du temps. Pendant trois, quatre ans, nous n'avons rien publié. Le temps se révèle donc une nécessité, une permanence. Nous le constatons encore aujourd'hui au travers de la recherche d'un vaccin contre la covid-19, et ce malgré les formidables progrès technologiques et les investissements massifs opérés par les États et les laboratoires. Le processus qui conduit à la découverte est bien davantage assimilable au feu qui prend lentement qu'à l'étincelle qui crépite soudainement. En ce sens, l'exercice de la programmation pluriannuelle sied parfaitement au domaine de la recherche. Les moyen et long termes lui sont constitutifs, et les chercheurs ont besoin de ce temps précieux, de cette visibilité pour avancer sereinement. Avoir du temps ne signifie en aucun cas avancer lentement. Au contraire, des conditions de recherche apaisées sont un gage de réussite. C'est sous cet angle que nous aborderons le projet de loi que vous nous soumettez, madame la ministre : offre-t-il des conditions satisfaisantes et ouvre-t-il des perspectives favorables à la recherche de demain ? Disons-le d'emblée, la réponse tend clairement vers la négative. Si nous nous réjouissions d'examiner ce texte tant attendu, étant tout à fait conscients du sous-financement chronique de la recherche depuis des années, nos motifs de satisfaction s'arrêtent ici. Tout d'abord, un hiatus entre la présentation de l'effort budgétaire qui serait réalisé par l'État sur la période 2021-2030 et la réalité des chiffres est important. Autrement dit, l'écart entre votre communication gouvernementale et les actes concrets pour la recherche est pour le moins étonnant. Je n'épiloguerai pas, mais cette loi de programmation manque doublement de sincérité et de crédibilité : d'abord, sur les montants déployés, qui ont été présentés avantageusement, mais qui restent- nombre de mes collègues l'ont dit -en deçà des enjeux actuels sur la période retenue, presque une décennie, durée jugée anormalement longue par le Conseil d'État, mais qui permet de reporter les investissements à plus tard, rendant par là même ceux-ci hypothétiques. Heureusement, notre commission est revenue, à la quasi-unanimité, à une forme de raison, en raccourcissant la période de programmation, dont le terme est désormais 2027, et en intensifiant l'effort budgétaire sur les premières années afin de répondre aux besoins urgents du monde de la recherche. Si vous tenez tant à relancer la recherche, comme vous le soutenez, portez réellement cette ambition et acceptez d'endosser maintenant la majeure partie de cet investissement, plutôt que de le renvoyer à un futur incertain

La déception et le rejet sont à la mesure de l'attente de la communauté. À l'image des votes du Cneser- je ne parle pas du vote final -, très majoritairement contre les dispositifs créés par ce projet de loi, des diverses motions votées dans les laboratoires et les universités, la communauté des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des vacataires et de l'enseignement supérieur ne vous suit pas. Votre communauté, madame la ministre, ne vous suit pas dans l'orientation de votre programmation. programmation. Avez-vous conscience de l'intensité du rejet que provoque votre texte ? Ce rejet n'est pas dogmatique ; il est étayé, argumenté. Notre groupe partage deux préoccupations fondamentales largement exprimées par cette communauté l'accentuation de la précarisation et le déséquilibre de notre modèle de recherche, qui devient trop axé sur la recherche sur projets. Sur le premier point, nous ne nous opposerons pas, par principe, à tous les contrats nouvellement établis. Le contrat postdoctoral comble un vide juridique et répond à une problématique précise d'inadéquation entre les contrats de travail existants et le recrutement des postdoctorants. Il constitue donc une avancée. Néanmoins, pour qu'il s'agisse d'une avancée, encore faut-il que cette batterie de contrats soit conforme à votre promesse, qui est aussi la nôtre, de lutter contre la précarité croissante attachée aux contrats des doctorants-chercheurs, et de leur garantir une rémunération à la hauteur du niveau de leur qualification et de leur engagement. Or c'est précisément à cet endroit que le bât blesse. Pour plusieurs d'entre eux, notamment les contrats doctoraux de droit public et de droit privé, ni durée ni rémunération minimales ne sont garanties ; et s'agissant du CDI de mission scientifique, nous sommes dans un « juridique ». Reconnaissez, madame la ministre, qu'en termes de protection des doctorants-chercheurs, nous pouvons faire mieux.

comment voulez-vous que notre recherche prospère quand les principaux concernés ont des contrats d'un an et doivent, au bout de six mois, se mettre à chercher un autre poste, une autre mission ? C'est impossible ! La stabilité est une condition du succès de notre recherche, pour l'unique et bonne raison invoquée dans mon introduction : le temps en la matière est indispensable. Il s'agit non pas de parti pris, mais simplement de bon sens. De manière analogue, la précarisation des doctorants chercheurs fait écho à la précarisation de notre modèle de recherche, résultant de la part excessive que représente la recherche sur projets. Nous ne disons pas qu'il faut mettre fin à la recherche sur projets. Nous estimons simplement qu'il convient de rééquilibrer notre modèle de recherche publique au profit du financement récurrent

D'ailleurs, rien ne prouve que la mise en concurrence à outrance par le truchement des appels à projets nourrisse véritablement la recherche fondamentale et les innovations de rupture, bien au contraire ... Enfin, j'aimerais aborder un « silence » de ce projet de loi qui, dans une certaine mesure, illustre la vision qui sous-tend cette loi de programmation : il s'agit de l'absence de continuum entre l'enseignement supérieur et la recherche ou, énoncé autrement, de l'absence d'une vision territorialisée de la recherche dans une logique d'aménagement du territoire. Historiquement, l'enseignement supérieur et la recherche ont fait partie intégrante de la réflexion et du processus d'aménagement des territoires. Or le postulat qui fonde cette loi de programmation, à savoir le déclassement de la recherche et de l'université françaises sur le plan international, accréditerait pour certains la thèse selon laquelle il est impératif d'avoir des établissements de taille critique pour rivaliser au niveau mondial. Dans cette perspective, il s'avérerait pertinent de concentrer l'essentiel des ressources sur quelques établissements. d'avoir des pôles d'excellence peut être bénéfique, bien sûr, et utile, sûrement, la concentration excessive des moyens sur quelques-uns se révèle pernicieuse à un triple titre. Premièrement, le rapport entre concentration des moyens dévolus à la recherche et production scientifique n'est pas solidement démontré à ce jour. Il s'agit davantage d'une position théorique que d'un constat ancré. Deuxièmement, ce modèle tend à effacer les logiques de coopération au seul profit des logiques de compétition, oubliant que la recherche a beaucoup progressé grâce aux activités menées en commun. Enfin, il ne prend aucunement en considération la problématique de l'organisation spatiale et, partant, celle du développement équilibré et dynamique de nos territoires. En d'autres termes, ce modèle va à l'encontre du mouvement de décentralisation et d'une attention accrue portée aux territoires. À cet égard, il est révélateur que ce soit notre commission qui ait corrigé cet oubli, en replaçant les collectivités territoriales au coeur du processus. J'aurais pu me féliciter d'intégrité scientifique- nous allons en parler -et dénoncer le recours aux ordonnances sur des sujets majeurs. Vous l'aurez compris, madame la ministre, il faudrait un grand miracle pour que nous puissions voter votre loi de programmation. Néanmoins, comme aiment à le raconter certains chercheurs, les découvertes sont parfois le fruit du hasard. Alors, sait-on jamais ! La

« la science n'est pas fille du seul étonnement et du désir de savoir » écrivait Jacques Blamont. Elle dépend aussi de la volonté des autorités et de l'environnement propice des institutions. Le Gouvernement a pris la mesure du déclin de la France en matière de recherche, et nous saluons cette initiative opportune ; celle-ci arrive après un long silence de près de quinze ans, durant lequel la France n'a bénéficié d'aucune loi de programmation pour la recherche. La valorisation des rémunérations et la mobilité des carrières sont des facteurs essentiels pour accroître l'attractivité des métiers à l'égard non seulement des talents étrangers, mais également de nos propres talents, de plus en plus tentés de quitter la France pour démarrer leur vie professionnelle dans de meilleures conditions. Dans de nombreux domaines tels que l'intelligence artificielle, la pénurie de compétences compromet nos perspectives industrielles et représente un handicap compétitif certain face aux champions mondiaux que sont les États-Unis, la Chine ou encore le Royaume-Uni. La cybersécurité fait aussi face à des pénuries constantes de talents, et nos entreprises, nos collectivités, nos administrations sont touchées de plein fouet par des attaques recrudescentes. Je pourrais également prendre l'exemple de la recherche biologique et médicale, bureaucratisée à l'excès et dévalorisée. Les meilleurs chercheurs émigrent pour rejoindre Harvard, Princeton ou Dallas, tandis qu'un désert scientifique se dessine peu à peu en France, au gré d'une lente dérive du financement de la recherche. Nous soutenons le raccourcissement de la durée de la loi de programmation à sept ans, comme l'ont acté conjointement la commission de la culture et la commission des finances. La dernière loi de programmation date de 2006 et n'a jamais été appliquée. La recherche française n'a plus le temps d'attendre. Nous devons aussi répondre au désarroi de milliers de jeunes chercheurs au déroulement de carrière indigne, privés de reconnaissance. J'aimerais insister sur l'impérieuse nécessité de redonner à la recherche fondamentale des moyens à la hauteur de ses besoins. Nous devons aussi nous méfier de l'hypercentralisation des infrastructures et des équipes. Il ne faudrait pas que la réforme du préciput, prévue à l'article 12, renforce les déséquilibres entre les territoires. Dans ce domaine plus que dans tout autre, les logiques de proximité, de mise en réseau et de coopération sont les plus fertiles. Il nous faut reconnaître la valeur des petites équipes, des petites formations, des jeunes chercheurs, qui ont beaucoup à proposer. La science procède souvent par rupture dogmatique avec les anciens. Elle se nourrit d'audace et d'idées nouvelles. Toute logique de reproduction du cadre dogmatique majoritaire l'étouffe, comme le décrit avec une grande lucidité Alexandre Grothendieck, génie des mathématiques, dans son autobiographie. Avec une immense générosité, il a soulevé des pans entiers d'une nouvelle connaissance jusque-là invisible, laissant derrière lui une oeuvre de 60 000 travaux, aujourd'hui supports d'intenses recherches. Il suffit parfois d'une personne, d'un regard nouveau posé sur des phénomènes anciens, pour renverser tout ce que nous savons ou croyons savoir. La recherche est avant tout l'art des humbles, de ceux qui n'ont pas peur de l'erreur, pour ne jamais dépendre des anciennes vérités dressées comme des dogmes contre une connaissance sans cesse renouvelée. François Jacob n'aurait sans doute pas révolutionné la génétique sans l'Institut Pasteur. Un cadre et des moyens sont nécessaires pour permettre aux 300 000 chercheurs de France d'aller au-devant des découvertes, avec toutes les incertitudes, les fulgurances, les reculs, les réveils, la persévérance que demande ce travail de l'ombre. Nous, sénateurs, députés, ministres,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce moment de crise sanitaire et climatique nous révèle au grand jour à quel point il est indispensable de donner les moyens nécessaires à la recherche publique. Ce n'est qu'avec des moyens ambitieux que notre pays pourra rester à la pointe de la recherche mondiale et contribuer à répondre à ces enjeux. C'est l'essence même de ce projet de loi qui affiche, du moins en théorie, le souhait de retrouver l'ambition de notre pays pour son système de recherche publique et de mieux accueillir la nouvelle génération de jeunes scientifiques, qui aura vocation à porter l'avenir de la recherche publique française. La communauté des chercheurs attendait énormément de ce projet de loi. L'enseignement supérieur souffre d'un manque criant d'investissements : l'effort de recherche publique n'a cessé de baisser depuis les années 1990. Alors que le nombre d'étudiants est en constante d'augmentation, de 14 % entre 2010 et 2017, le nombre d'enseignants, lui, est resté constant. Le personnel de l'enseignement supérieur connaît une forte précarisation : toujours plus de vacataires et de contractuels, toujours moins d'ouvertures de poste de titulaire, toujours moins de perspectives professionnelles pour les jeunes chercheurs. Cette précarisation est également due au manque de revalorisation des salaires des enseignants et des chercheurs, très au-dessous de la moyenne des pays développés. À cette précarisation s'ajoute l'insécurité permanente des financements, avec une proportion croissante des financements par appels à projets, par rapport aux crédits récurrents, c'est-à-dire les financements pérennes. Les chercheurs nous alertent en masse sur ce point : les appels à projets sont un bon complément des financements récurrents, mais ne doivent en aucun cas les remplacer. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés au point absurde où nous payons nos meilleurs chercheurs essentiellement pour qu'ils remplissent des demandes de financement et des rapports d'activité. Aussi, nous aurions espéré un projet ambitieux qui réponde à toutes ces attentes. Malheureusement, le projet de loi, en l'état, ne répond pas aux manques des universités et de la recherche publique française. Mes collègues du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires et moi-même regrettons son manque d'ambition financière, notamment sur les premières années. Malgré l'adoption en commission d'une programmation financière resserrée sur sept ans, le budget reste trop faible. Avec les projections d'inflation, il ne permettra pas d'atteindre l'objectif de la France d'investir un minimum de 3 % de sa richesse nationale dans la recherche. Nous sommes bien loin du minimum vital qui donnerait les moyens d'assurer un fonctionnement digne du service public de l'université. Pis encore, au lieu de pallier la précarisation que connaissent déjà les personnels de l'enseignement supérieur, ce projet de loi pour la recherche l'accentue avec la création des chaires de professeur junior et des CDI de mission scientifique, mais aussi avec l'absence de revalorisation salariale concrète et d'ouvertures suffisantes de postes. La philosophie de ce projet de loi est fondamentalement problématique, car il promeut un esprit de compétition entre les universités, notamment en valorisant encore davantage la logique des appels à projets pour l'obtention des financements. Cela a pour conséquence- nous l'avons vu -d'accentuer les inégalités entre structures et entre territoires, de favoriser les grandes universités, de gâcher des talents, de manquer des opportunités, et de plonger les personnels dans l'insécurité et le découragement. Il n'est donc pas étonnant que ce projet de loi, en complet décalage avec les attentes des acteurs concernés, ait suscité un rejet profond depuis plusieurs mois. Nous soutenons pleinement les revendications portées dans la pétition en faveur d'une autre loi pour la recherche, qui a déjà rassemblé plus de 20 000 signatures. Ce texte mérite d'être véritablement revu, pour proposer une loi de programmation de la recherche digne de ce nom, qui réponde aux attentes et prévoie des financements à la hauteur des enjeux. Investir dans la recherche est une décision politique, courageuse, essentielle. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires s'oppose donc à ce projet de loi en l'état actuel et dénonce son manque d'ambition. La parole

mes chers collègues, je remercie le groupe du RDSE, qui me fait le grand honneur de parler en son nom d'un sujet aussi fondamental que la recherche pour ma première prise de parole dans notre hémicycle. On peut être le plus vieux groupe parlementaire du Sénat et garder comme priorité l'avenir et les promesses d'amélioration de l'homme et de la société. C'est bien le but ultime de la recherche. J'en profite pour rendre hommage au sénateur Laffitte qui a présidé notre groupe et que vous avez dû connaître, madame la ministre, à Sophia-Antipolis. Il nous oblige. La richesse de la France est sa ressource humaine et l'intelligence de ses habitants. L'investissement primordial de notre société doit bien redevenir l'éducation de nos concitoyens et la recherche, qui en est l'aboutissement suprême. Je découvre que la procédure accélérée a été mise en oeuvre pour l'adoption de ce projet de loi, certainement censée appuyer l'urgence qu'il y a à agir pour la recherche et tous ceux qui la font. Nous mesurons tous le décrochage de la France par rapport aux autres pays de l'OCDE ces dernières années. Plusieurs facteurs en sont responsables : sous-investissement chronique, baisse de l'attractivité des carrières scientifiques, découragement dans les laboratoires, rigidités des outils de gestion des organismes de recherche, insuffisances des passerelles entre le public et le privé. Les défis sont nombreux et ce projet de loi doit ramener la France parmi les nations leaders en matière d'innovation technologique, et ainsi améliorer sa place dans les classements internationaux. Pour cela, on nous annonce 25 milliards d'euros de crédits nouveaux sur dix ans, l'objectif étant de parvenir, par effet de levier sur la recherche privée, à la cible de 3 % du PIB à l'horizon 2030, dont 1 % de financement public. Cela passe par une importante mobilisation et de fortes synergies entre public et privé. Notre groupe salue cette trajectoire ambitieuse, dans un cadre budgétaire contraint. Cette loi donne à la communauté scientifique une perspective sur le long terme, afin d'assurer aux équipes de recherche des niveaux de crédits et de moyens humains sur un temps plus long, qui correspond davantage au temps de la recherche que celui d'un exercice budgétaire. Cependant, si dix ans peuvent donner une impression, ou une illusion, de pérennité, sept années seulement permettent d'allier besoin de sécurité et réalisme budgétaire. La visibilité ainsi donnée à nos universités et à nos organismes de recherche doit permettre de lutter contre la fuite des cerveaux. Si la recherche est universelle et les échanges internationaux profitables, trop nombreux sont les départs définitifs de nos plus brillants talents

Nous nous inscrivons dans un temps suffisamment long avec des enjeux essentiels. Nous devons réussir plusieurs grandes transitions : celle de l'écologie, celle du numérique. Le monde de la recherche sera un acteur décisif pour faire face aux enjeux primordiaux dans les domaines des énergies propres ou de l'intelligence artificielle, aux côtés des enjeux sanitaires et alimentaires. Cette loi doit aussi concilier protection des chercheurs et souplesse en faveur des organismes de recherche. Enfin, elle procède à une revalorisation salariale des métiers de la recherche en imposant un seuil de deux SMIC pour l'embauche des jeunes chercheurs. Notre groupe est sensible à l'attention portée à l'attractivité des carrières scientifiques, alors que le nombre de doctorants est à la baisse. Beaucoup reste à faire pour sensibiliser nos plus jeunes, et particulièrement les jeunes filles, aux carrières scientifiques. Le projet de loi crée deux nouveaux dispositifs- la chaire de professeur junior et le contrat postdoctoral -, qui doivent permettre d'accroître l'attractivité et de favoriser les synergies entre privé et public. Ce peut être un levier important de souplesse des outils de gestion des ressources humaines pour les organismes de recherche, qui pourront mieux s'adapter aux contraintes des projets de recherche. Ainsi, 1 400 chaires de professeur junior pourront être créées, dans des domaines nouvellement explorés. L'Assemblée nationale a réduit de 25 % à 20 % la limite des recrutements autorisés pour ces chaires. Je ne pense pas que le Sénat doit se sentir obligé d'aller plus loin en réduisant encore cette limite. Cette innovation nous offre une chance de faire des recrutements atypiques dont la recherche a aussi besoin. Originaire du Beaujolais, à côté de la maison natale de Claude Bernard, je suis forcément influencé par cet immense savant devenu professeur au Collège de France, malgré son échec au baccalauréat. Ce texte prévoit enfin de lutter contre la complexité des procédures et de donner un nouveau souffle à la coordination entre universités, organismes de recherche publics et privés, et monde de l'entreprise. Car s'il est un domaine où nous excellons en France et dans lequel il faut cesser toute recherche, c'est bien celui de la complexité administrative, domaine dans lequel J'espère que ce projet de loi permettra à la politique publique de la recherche de se doter d'une orientation claire et ambitieuse en faveur de notre communauté scientifique et d'associer les collectivités territoriales pour favoriser ces espaces de brassage intellectuel indispensables à l'émergence de nouvelles connaissances. Tel est l'esprit qui sous-tend nos contributions pour enrichir ce projet de loi.

Ce décrochage a des conséquences en termes de souveraineté- toutes celles et tous ceux qui sont attachés à la souveraineté industrielle et économique de la France savent

de l'état des savoirs et des connaissances, et non pour divulguer telle ou telle idéologie, quelle qu'elle soit. Enfin, nous aurons un débat sur les territoires- la commission a fait un travail intéressant -ou sur ce qu'est l'excellence à la française.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le 19 mars dernier, le Président de la République annonçait pour la recherche un effort budgétaire inédit depuis la période de l'après-guerre. Pourtant, de l'après-guerre. Pourtant, le CESE a émis, à l'unanimité, un avis négatif sur la présente loi de programmation. Avec la même unanimité, les présidentes et présidents des 46 sections et commissions du Comité national de la recherche scientifique et des dix conseils scientifiques des instituts du CNRS ont

Enfin, les organisations syndicales nous ont toutes exprimé leur opposition à ce texte, y compris celles qui ont signé avec votre ministère le protocole d'accord sur les revalorisations. Pourquoi une telle ingratitude alors qu'une manne, d'une générosité quasi biblique, viendrait secourir et revigorer la recherche publique comme jamais depuis la Libération ? « On ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens », disait le cardinal de Retz. Les hyperboles amphigouriques passées, il reste la terrible réalité des chiffres. Notre commission des finances, à la suite d'un travail de déconstruction critique exemplaire, nous le montre : selon les projections réalisées, « sur le périmètre de la loi de programmation [ ...], la trajectoire retenue se borne à stabiliser la part des dépenses de recherche dans le PIB ».

rapporteur, Jean-François Rapin, dont je salue la qualité du travail, ajoute que « la France ne pourra conserver son rang de grande puissance scientifique qu'au prix d'un effort budgétaire sans précédent ». gouvernement auquel vous appartenez abandonne l'objectif de porter notre effort de recherche à un niveau équivalent à celui de nos homologues européens, mais, de plus, la présente programmation consacre le renoncement à l'ambition ancienne et toujours réaffirmée d'atteindre le ratio mythique des 3 % du PIB pour la recherche. Le 7 septembre dernier, sur le campus de l'Université Paris-Saclay, le Premier ministre déclarait Je vous mets au défi de trouver une période, depuis 1945, où l'État a décidé volontairement de dégager autant de moyens. » La chose est aisée Le 14 février 1959, à Toulouse, le général de Gaulle déclare : « L'État [ ...] a le devoir d'entretenir dans la Nation un climat favorable à la Recherche et à l'Enseignement. Son gouvernement met en oeuvre rapidement cet engagement et le budget du CNRS, qui est de 8 milliards de francs en 1958, est porté à plus de 15 milliards en 1960, soit un quasi-doublement en deux ans. Cette distorsion terrible entre les annonces gouvernementales, ainsi que la faiblesse du croît budgétaire porté par ce projet de loi, est vécue par la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche comme une humiliation supplémentaire, car elle vit quotidiennement la lente, mais inexorable dégradation de ses conditions de recherche et d'enseignement. Je pense tout particulièrement à celles et à ceux sans lesquels tout notre système aurait déjà sombré et dont la seule perspective de carrière est d'enchaîner les contrats jusqu'à la retraite. Sans doute près de la moitié du volume des travaux réalisés dans le cadre du service public de la recherche et de l'enseignement est assurée par ces salariés contractuels.

il ressort le sentiment qu'il a été conçu par et pour une poignée d'établissements dont les premières places au classement de Shanghai constituent l'unique objectif. Vous nous permettrez de ne pas partager ses critères d'évaluations conçus par le parti communiste chinois et de continuer de défendre l'idéal républicain d'une science au service de la Nation apprenante, de l'émancipation humaine, de l'exercice de la critique et de la recherche perpétuelle de la vérité comme seule vérité. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, face aux incommensurables défis que notre monde complexe soumet jour après jour à l'esprit humain, face en particulier aux périls qui nous menacent aujourd'hui, sans recherche, point de salut ! Point de salut économique, puisque seule l'innovation peut nous permettre de survivre dans un monde régi par le numérique et les biotechnologies. Point de salut environnemental non plus pour réussir la transition énergétique. Nous ne pouvons donc que souscrire à l'objectif de la présente loi de programmation. Il faut augmenter l'effort de recherche de la Nation. Les 3 % du PIB, correspondant à l'engagement de Lisbonne, ne sont pas un fétiche ; ils constituent notre balise. La présente loi de programmation permettra-t-elle d'atteindre cet objectif ? C'est là que les choses se compliquent, car on ne peut pas vraiment le savoir. Ce texte est trop ciblé pour nous permettre d'en avoir le coeur net. Il ne porte en effet que sur une partie de l'effort public. La recherche privée est exclue du champ de cette loi de programmation. C'est un vrai problème pour avoir une vue d'ensemble du dispositif, puisque la recherche privée représente les deux tiers de l'effort de recherche du pays. C'est sur elle que repose principalement l'objectif des 3 % du PIB, puisqu'elle est censée atteindre 2 % de celui-ci d'ici à 2030. La recherche privée se fonde pour sa plus grande part sur le crédit d'impôt recherche, le CIR, qui n'est malheureusement pas traité dans le présent texte. Techniquement, le CIR étant un dispositif fiscal, il ne peut être réformé que dans le budget. Mais il nous manque au moins un schéma d'évolution prospective de son impact sur l'effort de recherche privée.

L'effet de levier paraît d'autant plus hypothétique et compromis que, parallèlement à la loi de programmation pour la recherche, le projet de loi de finances pour 2021 réduit la voilure du CIR. Dans ces conditions, l'objectif des 3 % n'est-il pas d'emblée inatteignable ? On ne peut pas prétendre relancer l'effort de recherche sans s'interroger sur le CIR, en particulier sur le décalage entre sa générosité et son impact sur le niveau de recherche privée. En comptant sur l'effet de levier entre le public et le privé, la LPPR se concentre donc sur la dépense publique, ou plutôt sur la seule dépense publique d'État- et encore, pas totalement.

concernés. donc les crédits des établissements de recherche rattachés aux ministères de l'économie, de la transition écologique et de l'agriculture. La recherche et développement de la défense ne figure pas non plus dans la trajectoire. Un cinquième des crédits publics d'État sont donc hors LPPR. Par ailleurs, ni les crédits de recherche des collectivités, ni les crédits européens, ni ceux du plan de relance et du programme d'investissement d'avenir ne sont pris en compte. Nous défendrons un amendement pour qu'ils le soient. Car, en l'état actuel des choses, l'ensemble de l'effort public de recherche n'apparaît pas clairement. Il était par ailleurs compromis par la longueur de la programmation envisagée par le Gouvernement. Sur dix ans, l'inflation conduit à absorber la quasi-totalité de l'augmentation prévisionnelle des crédits. Nous nous réjouissons donc que notre commission, sous la houlette de notre excellente rapporteure, Laure Darcos, ait réduit la durée de la programmation à sept ans. L'effort est désormais plus tangible. Il faut cependant se garder de réduire le débat à l'aspect quantitatif des choses. La répartition des crédits sur le territoire compte aussi. Pour éviter d'accentuer la concentration des crédits, le Gouvernement a choisi de les faire passer par l'Agence nationale de la recherche plutôt que de les allouer directement aux pôles universitaires. Nous comprenons bien la stratégie, mais quelle garantie que cela porte ses fruits ? Comme vous le savez, madame la ministre, nous avons été destinataires de nombre de remontées de terrain faisant état de la crainte inverse, qui ne semble pas infondée. En effet, pour répondre à un appel d'offres de l'Agence nationale de la recherche, il est évident que les grands pôles universitaires sont mieux équipés. Pour éviter cet écueil, nous défendrons un amendement imposant à l'Agence nationale de la recherche de prendre en compte la dimension territoriale de la répartition de ces crédits. Ce n'est pas non plus un texte sur l'université et, là encore, c'est bien dommage, parce qu'il est assez artificiel de séparer les laboratoires de l'ensemble de l'écosystème de l'enseignement supérieur. L'université doit être réformée, madame la ministre. Elle ne l'a pas été depuis la loi Pécresse de 2008. Il faut, par exemple, briser le tabou de la sélection pour l'entrée en licence. Cette problématique de l'excellence de l'université est directement liée à celle de la recherche, car une université plus performante est aussi une université qui coûtera moins cher et dont les crédits économisés pourront être affectés aux laboratoires de recherche. C'est une question de philosophie générale, qui traduit à nos yeux l'étroitesse du périmètre de la LPPR. Sous réserve de ces observations, et compte tenu des modifications apportées au texte en commission, vous l'aurez compris, madame la ministre, le groupe centriste aborde cette discussion sans opposition de principe. Nous espérons juste que certains amendements

Il y a incontestablement un large consensus pour convenir de la dimension stratégique lorsqu'on évoque les missions de notre défense nationale, mais cela semble beaucoup moins évident lorsqu'on fait référence à notre recherche. Pourtant, s'il ne fallait prendre que ce seul exemple, la violence de la crise sanitaire que nous traversons, avec son lot de questionnements et d'espoirs scientifiques, renforce, si besoin était, la nécessité d'une recherche à la hauteur des enjeux contemporains. S'inscrivant dans le temps long, les travaux de nos chercheurs portent en effet l'espoir de répondre à des transformations profondes de notre société, comme la transition énergétique ou l'intelligence artificielle. L'opinion publique en a sans doute une perception partielle et diffuse, alors que c'est fondamental pour notre avenir. le temps de gestation particulièrement long de cette loi de programmation de la recherche n'est sans doute pas étranger à l'intensité des attentes qu'elle suscite ni à l'ampleur des manifestations hostiles à son encontre. Très sincèrement, pour avoir participé aux auditions menées par notre rapporteure Laure Darcos, je dois admettre que la synthèse objective des avis enregistrés relève de la gageure. J'en profite pour saluer le travail de qualité réalisé par ma collègue rapporteure, dans des conditions très défavorables à un examen parlementaire éclairé, puisqu'elle l'a réalisé dans des délais plus que contraints et en plein renouvellement sénatorial. Je remercie également nos administrateurs de la finesse de leur concours et de l'ampleur de leur disponibilité. Madame la ministre, mes chers collègues, de nombreux indicateurs font état d'un diagnostic sans appel, que nous partageons de manière unanime : la recherche française décroche. Son sous-financement chronique ne lui permet plus d'espérer figurer dans le peloton de tête des nations qui font avancer la science, et nos meilleurs talents comprennent vite qu'il leur faut quitter le territoire national pour mener à bien leurs travaux. L'itinéraire d'Emmanuelle Charpentier, lauréate cette année du prix Nobel de chimie, est éloquent : après un parcours académique exemplaire, c'est outre-Atlantique qu'elle a trouvé les financements nécessaires à l'éclosion de son talent. Le deuxième constat est celui d'un décalage entre les annonces du processus de Lisbonne en 2000 et la réalité de l'effort budgétaire réellement consenti, loin de l'objectif de 3 % du PIB consacré à la recherche. Dans le contexte actuel, on peut cyniquement observer que, à dépenses constantes, la baisse brutale de notre PIB cette année a mécaniquement fait monter ce taux d'effort. Mais là n'est évidemment pas l'objectif de cette LPPR. Consacrer davantage de moyens à la recherche, mieux armer l'Agence nationale pour que davantage de projets soient validés, donner de réelles perspectives sur le temps long : voilà ce qu'attend l'ensemble de la communauté scientifique. Madame la ministre, je ne doute pas un seul instant que ce soit également votre volonté, mais je dois d'abord vous faire part de ma déception concernant la présentation formelle de ce plan. J'ai naïvement tendance à croire que, lorsque les mesures sont sincères, il n'est nul besoin de les gonfler par un quelconque artifice de marketing. Hélas ! l'inhabituelle présentation des dépenses sous forme cumulative, largement pointée par le Conseil d'État, génère d'emblée une suspicion de programmation bodybuildée qui dégonflera rapidement. De plus, la quasi-concomitance de cette présentation avec les mesures du plan de relance et le début de l'examen du projet de loi de finances ne concourt pas à une extraordinaire lisibilité. Toutefois, le plus grave est ailleurs, avec la durée exceptionnellement longue de cette programmation. Se projeter dans dix ans, c'est vouloir engager la responsabilité des exécutifs des deux prochains quinquennats. Ce n'est pas sérieux ! La nette concentration des efforts sur les cinq dernières années de ce plan ajoute au discrédit et nuit gravement à l'ambition affichée avec force communication, tout en occultant le renoncement à l'objectif de financement à hauteur de 1 % du PIB de la recherche publique. Fort judicieusement, notre commission a décidé de revenir à un tempo plus cohérent, en inscrivant le texte dans un horizon de sept ans, ce qui correspond à la durée communément appliquée pour une loi de programmation. Je le dis comme je le pense, conserver cet agenda est un gage indispensable, que le Gouvernement doit collectivement accepter. Il y a un troisième constat, moins consensuel : la complexité et la rigidité de la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs, unique au monde. Avec les chaires de professeur junior (CPJ) et les contrats de mission, vous souhaitez, madame la ministre, ouvrir la voie à de nouveaux profils, comme nous avons pu le découvrir ensemble à Angers lors de votre récente visite ministérielle. Sur ce point, vous avez courageusement décidé de lever les freins, au risque de vous heurter à une large partie des représentants syndicaux, plus attachés à la défense de statuts que soucieux de se mettre en phase avec le monde qui bouge autour d'eux. J'interprète l'accord majoritaire obtenu à l'arraché il y a deux semaines comme la timide adhésion à un modèle modernisé auquel je veux bien croire, mais dont il n'a pas été fait la preuve de son absolue nécessité. Pour garantir que ces CPJ ne seront pas des voies expresses vers une titularisation à moindre exigence, j'ai fait adopter en commission un amendement pour exiger des futurs lauréats une habilitation à diriger des recherches en plus des garde-fous inscrits dans l'article 3. Enfin, en tant que rapporteur pour avis de la mission « Recherche et enseignement supérieur », permettez-moi de rappeler que les établissements d'enseignement supérieur et de recherche sont le premier opérateur public de recherche en France. Tutelle indispensable de nombreux projets, ils bénéficieront de davantage de lisibilité grâce à une meilleure définition du préciput. Mais nous devons aussi veiller à conserver leur visibilité auprès de tous les acteurs de la recherche. Comme vous tous, je suis convaincu que notre société devrait considérer davantage notre jeunesse, nos étudiants, nos docteurs et nos chercheurs. Il est indispensable pour cela d'investir dès maintenant, et de ne pas remettre à plus tard ce que l'état de notre recherche exige de nous aujourd'hui.

la Haute Assemblée va dépasser le temps présent pour regarder loin, et échanger durant cette semaine sur la recherche, c'est-à-dire l'avenir de notre pays, ardente obligation du plan.

insuffisamment systémique et structurante, de son propre aveu, même si elle n'est pas exempte d'avancées et de rattrapages bienvenus. Tout a été exprimé par nos trois excellents rapporteurs, Laure Darcos, Jean-François Rapin et Jean-Pierre Moga sur l'étalement de cette loi de programmation, qui allait dans sa version initiale au-delà de l'horizon des deux quinquennats que peut constitutionnellement exercer l'actuel chef de l'État. De manière pertinente, notre commission a ramené la projection à une durée habituelle de sept ans. C'est une bonne chose. Il semblerait d'ailleurs que le message du Sénat ait été entendu, au moins partiellement. Les projections du plan de relance pour les deux prochaines années ainsi qu'un amendement du Gouvernement corrigent, sinon la trajectoire initiale de la LPPR, du moins le péché initial qui était le sien.

De même, je veux saluer les efforts de revalorisation des régimes indemnitaires des chercheurs et enseignants-chercheurs, en particulier en début de carrière. Ils permettront de réaligner progressivement les grilles indiciaires sur la moyenne des pays de l'OCDE, ce qui est un minimum pour revaloriser le métier d'enseignant-chercheur et, espérons-le, pour renouer avec une attractivité perdue. Il était également important de trouver des solutions pour retenir les jeunes talents. Tous ne rêvent pas de carrières à l'ancienneté. Tous ne rêvent pas d'emplois à vie. Tous veulent disposer de contrats et de moyens diversifiés pour mener leurs travaux dans des conditions sécurisées. Je souhaite que les chaires de professeur junior répondent à leurs aspirations. Je sais et comprends l'attachement de la communauté scientifique aux concours statutaires de recrutement. Pour autant, oui, il faut répondre à des besoins spécifiques des établissements. Oui, il faut offrir à nos jeunes talents des solutions plus satisfaisantes que les montages actuels, peu attractifs et pourvoyeurs de précarité. Madame la ministre, malgré cette avancée, que je salue de nouveau, je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a plusieurs rendez-vous manqués, tout d'abord celui de la confiance et du consensus avec la communauté scientifique sur un horizon et un avenir ambitieux. Les enjeux de l'avenir auraient pu être davantage partagés. Ce n'est pas le cas. Rendez-vous manqué, ensuite, pour revaloriser le statut des doctorants et la place du plus haut niveau académique dans notre société et dans l'organisation de notre État. Faibles rémunérations, faible valorisation, le doctorat demeure dans l'ombre des concours et des diplômes des grandes écoles françaises. Sans revenir sur ces concours, qui participent également à construire la méritocratie républicaine, je crois qu'il nous faut réfléchir aux moyens de mieux les valoriser. Plusieurs amendements du Sénat, cher Stéphane Piednoir, vont en ce sens. Rendez-vous manqué, également, pour s'interroger sur le rôle de l'université en tant qu'institution majeure du territoire en matière de recherche et d'innovation. L'approche territoriale me semble une fois de plus avoir été ignorée. Permettez-moi de dire mon étonnement qu'un projet de loi de programmation, dont l'objectif est de replacer la recherche dans une relation ouverte avec la société, fasse aussi peu référence à l'ancrage et à la diffusion de la recherche dans les territoires et au partenariat avec les collectivités locales. L'effet métropolitain, si décrié, n'est-il pas une nouvelle fois à l'oeuvre ? Cette LPPR n'impacterait-elle pas négativement les capacités de recherche, d'innovation et d'enseignement supérieur des villes universitaires non métropolitaines ? La mise en réseau de la recherche nécessite une approche multiscalaire autrement plus fine. Je crains que la dynamique qui innerve cette LPPR ne se fasse au détriment des équilibres régionaux et territoriaux en matière d'aménagement du territoire. Rendez-vous manqué, enfin, au moins dans le texte initial, pour réaffirmer les libertés académiques, c'est-à-dire la garantie pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs de mener leurs activités pédagogiques et scientifiques en toute indépendance. Héritées du Moyen Âge, ces libertés ont construit une université libre dans ses recherches et dans sa parole. Elles sont aujourd'hui mises à l'épreuve par la diffusion d'une conception anglo-saxonne de l'université, empreinte de bien-pensance et d'autocensure. Je crois que vous êtes sensible à ce sujet, madame la ministre, vous qui aviez assisté à la représentation reprogrammée de la pièce d'Eschyle,, en Sorbonne, il y a deux ans, et qui avez livré au quotidien, cette semaine, une tribune attendue sur cette question. Au-delà de ces atteintes insupportables à la liberté d'expression, la préservation intransigeante des libertés académiques est le gage de l'excellence de la recherche française. Aussi, je souhaite qu'à l'occasion de l'examen de cette LPPR, nous puissions échanger sur ce sujet important dans les travaux quotidiens des chercheurs, des enseignants et des enseignants-chercheurs. Je sais, madame la rapporteure, que c'est aussi votre souhait. Je me réjouis par avance des débats que nous aurons et des apports du Sénat sur ce sujet qui touche à la liberté d'expression au coeur même de l'université. Elle en est, historiquement, le berceau et la garante, et nous en mesurons en ces temps troublés la précieuse valeur.

Le travail reste long, et nous avons ressenti, à travers les nombreux textes que nous avons reçus, combien l'impatience était grande et combien il était dommage que vous n'ayez pas su, à l'occasion de ce projet de loi, nouer le consensus, le dialogue et la confiance que la communauté scientifique était en droit d'attendre.

plan de relance consacrés à la recherche sur les deux prochaines années. Le choc que vous appelez de vos voeux, et que vous avez voulu traduire en raccourcissant la durée de la programmation et en augmentant les premières marches, a

seront consacrés, au travers du programme d'investissements d'avenir, au soutien à la recherche privée, hors plans aéronautique et automobile, qui disposent eux aussi

C'est la raison pour laquelle il est ici demandé de les inscrire enfin expressément dans la loi. À un moment particulier où nous voyons la liberté d'expression fondamentalement remise en cause dans notre pays, notamment dans l'enseignement, il serait bon d'adopter de manière consensuelle cet amendement pour réaffirmer notre attachement à ce principe pour tous les enseignants-chercheurs. Quel

jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires

Les libertés académiques caractérisent la liberté professionnelle réservée aux universitaires et aux chercheurs. Elles sont la condition d'existence de leur métier et par là même la condition d'existence du progrès des connaissances. Elles se déclinent principalement en trois volets : la liberté de recherche, la liberté d'enseignement et la liberté d'expression. Héritées de la tradition universitaire née au Moyen Âge et de l'esprit des Lumières, les libertés académiques ne sont plus en France à l'abri d'atteintes manifestes. Plusieurs exemples récents le prouvent, qu'il s'agisse de menaces proférées à l'encontre d'enseignants ou de chercheurs participant à des débats, d'intimidations d'intimidations visant le contenu de travaux de recherche, de violences verbales ou physiques perpétrées contre des enseignants. Le terrible drame survenu à Conflans-Sainte-Honorine montre plus que jamais la nécessité de préserver, au sein de la République, la liberté d'enseigner librement et de former les citoyens de demain. Dans ce contexte, il paraît indispensable de réaffirmer les libertés académiques et de les conforter dans la loi. L'indépendance et la liberté d'expression des enseignants, des enseignants-chercheurs et des chercheurs sont déjà reconnues à l'article L. 952-2 du code de l'éducation, issu de l'article 58 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, dite « loi Savary ». Aux termes de cet article, « les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité ». Le présent amendement vise à compléter cet article, en précisant que les libertés académiques s'exercent dans le respect des valeurs de la République. Il s'agit d'inscrire dans la loi que ces valeurs, au premier rang desquelles la laïcité, constituent le socle sur lequel reposent les libertés académiques et le cadre dans lequel elles s'expriment.

sur les règles de fonctionnement de la communauté scientifique et la façon dont elle peut se protéger des pressions extérieures. Je dois à cet

les droits des chercheurs et de réaffirmer les principes de liberté de la recherche et d'indépendance, mais aussi d'intégrité scientifique. Le monde de la recherche fait face à des dérives préoccupantes- risque accru de « malscience » ou « mauvaise science », course aux publications, conflits d'intérêts, procédures bâillons visant à intimider les chercheurs, etc. Cet amendement réaffirme l'obligation faite à chaque chercheur, enseignant ou enseignant-chercheur de respecter l'intégrité scientifique, mais il réaffirme aussi leur droit leur droit à bénéficier de conditions qui le permettent. Ainsi, les règles des établissements doivent garantir, en toute circonstance, la liberté d'expression, l'indépendance et la recherche de l'intégrité scientifique.

je ne suis pas à l'aise avec l'approche que proposent ces amendements, parce qu'ils semblent conditionner la liberté académique à l'intégrité scientifique et je ne voudrais pas que nous ayons un faux débat ou un débat mal posé, dans lequel l'intégrité scientifique serait vue comme une restriction à la liberté d'expression.

car la libre expression ne peut s'exprimer que dans le cadre d'un État de droit qui protège de la violence, à l'image des hommes d'armes qui déposaient leur arsenal avant d'entrer en Sorbonne.

les mêmes garanties que celles dont disposent par la loi les enseignants-chercheurs et d'assurer ainsi une cohérence légale

L. 411-3 du code de la recherche prévoit que l'autonomie de la démarche scientifique et la libre circulation des idées sont aussi des garanties fondamentales.

la liberté d'expression. Ce consensus montre bien que tout cela est intrinsèquement lié à la vision que nous avons de l'université et de l'enseignement supérieur en général. Cet amendement est très complémentaire des discussions que nous venons d'avoir et de l'amendement présenté par notre rapporteure, puisqu'il vise à faire appliquer cette liberté d'expression, notamment quand il existe une volonté délibérée de s'opposer à un débat non pas de manière contradictoire comme cela est souhaitable, mais

à celui de l'enseignement scolaire constitue en quelque sorte une diminution des libertés académiques, dont nous venons justement de défendre le principe. C'est pour cette raison que je préférerais que nous nous accordions sur l'amendement qui suit, à savoir le mien

au président, pour faire respecter l'ordre dans le campus comme il le souhaite. Cela me semble une meilleure garantie par rapport aux principes constitutionnels.

se trouve juste à côté d'ici. La charte de Philippe Auguste affirme : « Ni le prévôt, ni aucun magistrat n'arrêtera un écolier ni ne l'emprisonnera, à moins que l'énormité du délit n'oblige à une arrestation immédiate. »

l'avis du Gouvernement ?

si vous la comparez à une série d'autres dépenses, par exemple les dépenses d'allègements de cotisations sociales, dont on nous dit à longueur de journée qu'elles vont donner de l'attractivité à notre pays. je peux vous dire que, si la France ne redresse pas la barre du côté de la recherche et de l'innovation, son attractivité ne va faire que décliner ! Ce n'est pas une simple aide à la baisse du « coût du travail »

Je vais oser un propos un peu décalé, peut-être pas très académique, mais nous sommes au début de l'examen du texte, et j'avais envie de m'exprimer ainsi. On va beaucoup parler de recherche, de science et, partant, de progrès. Notre société moderne est une société dite « de progrès ». Jamais nous n'aurons connu autant d'avancées, et la recherche scientifique y a apporté une immense contribution, mais il n'aura pas fallu plus d'un demi-siècle à la science pour mettre la planète au bord du gouffre et la vie humaine en péril. Pourtant, des scientifiques, très tôt, avaient

le croisement de l'ensemble des sciences au service d'un véritable progrès, pour en finir avec la science unique, au service d'une pensée unique, pour un modèle unique. En cette période trouble, dans ce monde insensé en quête de sens, au-delà de la science, réhabilitons aussi le rôle de la poésie, pour un progrès où science rime avec conscience et politique avec éthique.

regardons tout de même d'où nous venons ! On l'a plus ou moins tous dit dans la discussion générale : il y a eu une baisse de 40 % des crédits de l'Agence nationale de la recherche entre 2010 et 2015 ; nous n'avons pas respecté l'objectif de Lisbonne depuis quinze ans. On ne peut pas reprocher à un texte

braquet », j'aurais aimé que tout le monde le soit ! Les 6,5 milliards d'euros du plan de relance, avec un programme prioritaire de recherche lancé chaque mois,

une ambition budgétaire, confirmée dans le plan de relance, c'est aussi penser à l'avenir dans une période de crise et de pessimisme. C'est être capable de voir un cran plus loin, en soutenant la recherche. C'est extrêmement important à mes yeux. Comme tout le monde veut soutenir la recherche, je n'ai vraiment aucun doute sur le fait que, à chaque clause de revoyure, tous les trois ans, vous augmenterez ce budget de la loi de programmation ... Croyez-moi, j'en serai ravie, où que je sois